Monsieur le Premier ministre, lors de votre déclaration de politique générale, vous avez décidé de hurler avec les loups en évoquant une « écologie de la brutalité

c’est celui des industriels, qui ont changé leurs modes de production ; celui des agriculteurs, qui ont fait des efforts en matière de conversion ; celui de toute une société qui se mobilise pour défendre la planète.

pour permettre à notre pays d’avancer. Je vous confirme que nous ne nous livrerons pas à une opposition entre ruraux et urbains,… Nous non plus ! … entre les Français qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, ou tout simplement pour vivre, et les Français qui peuvent s’en passer, entre les agriculteurs et la planète. Je n’accepterai jamais les discours… Et les actes ? … qui visent en permanence à culpabiliser, à punir, à sanctionner, à brutaliser. L’écologie à laquelle je crois – et vous devez aussi le respecter – est une écologie qui

Monsieur le Premier ministre, le clivage, c’est vous ! Ce que je vous reproche, c’est la brutalité de votre immobilisme Jean René, 50 ans, est décédé dans les Côtes d’Armor après avoir respiré le sulfure d’hydrogène émis par les algues vertes lors d’un jogging : brutal ! Théo, 16 ans, a subi cinquante quatre interventions sous anesthésie générale pour reconstruire ses systèmes digestif et respiratoire. Une bataille de chaque instant pour respirer, manger et parler. Le glyphosate en est le responsable avéré : brutal ! Marie, apicultrice bio dans le Trièves, voit ses abeilles disparaître année après année, avec un taux de mortalité de 35 %. Les pesticides sont la première cause brutal ! Marius, agriculteur dans l’Anjou, ne peut plus consommer l’eau de son robinet, polluée par des solvants : brutal ! Noémie, en Guadeloupe, veut un enfant. Elle sait cependant que le chlordécone, trente ans après son interdiction, affectera le cerveau de son bébé brutal ! Lucas, 6 mois, issu d’une famille modeste habitant au bord du périphérique, a été hospitalisé en urgence pour une bronchiolite sévère due à la pollution : brutal ! Cette brutalité, ces punitions aveugles, cette décroissance du vivant, cette injustice érigée en dogme entre ceux qui peuvent tout et ceux qui subissent, c’est votre bilan. Voilà la brutalité ! Et la brutalité, c’est votre renoncement

sur le plan de l’attractivité et de la fidélisation des personnels soignants. Ces difficultés sont liées à plusieurs facteurs externes, bien identifiés, sur lesquels les établissements n’ont pas de prise. Le déficit est évalué à 1,2 milliard d’euros à la

locaux et une fragilisation profonde des opérations d’investissement. Des mesures d’urgence, monsieur le Premier ministre, permettront sûrement de rectifier cette tendance négative. De plus, la mise en place d’une stratégie de financement à long terme, pour continuer à investir, innover et soigner

Monsieur le Premier ministre, allez vous activer tous les leviers nécessaires pour aider nos établissements de soins à évoluer avec sérénité ? La

attache à la santé, particulièrement à l’hôpital. La semaine dernière, dans son discours de politique générale, M. le Premier ministre a rappelé combien l’hôpital était notre joyau.

par les élus, puisque ce sont les maires qui président les conseils de surveillance des établissements. Je partage en grande partie vos propos, en particulier sur le rôle de l’hôpital dans notre pays, l’implication des personnels et le retour

remercie, madame la ministre, pour cette réponse qui me convient parfaitement. Vous appliquez ici une règle que j’aime beaucoup : les amours, c’est bien ; les preuves d’amour, c’est mieux !

Monsieur le ministre, nous partageons tous ici une conviction : l’agriculture est constitutive de notre identité. Nous sommes fiers de nos agriculteurs, de leur engagement passionné, et nous ne pouvons qu’être à l’écoute de leurs revendications légitimes. Dans mon département du Haut Rhin, j’ai rencontré, comme chacun d’entre nous, de nombreux agriculteurs qui m’ont fait part de leurs difficultés, et surtout de leur sentiment de ne pas être entendus. Freins administratifs, concurrence déloyale et surtout faiblesse de leurs revenus… Tel est le ras le bol qu’ils ont exprimé. En trente ans, ce revenu a chuté de 40 % en France, bien loin de refléter les efforts, la passion et le travail qu’ils fournissent au quotidien. Avec les lois Égalim 1 et 2, que le Gouvernement a courageusement portées, nous avons répondu à une partie des inquiétudes de nos agriculteurs en inversant la construction du prix. Cependant, l’application de ces textes n’est pas satisfaisante. Monsieur le ministre, mon groupe a accueilli avec satisfaction l’annonce du doublement des contrôles que votre administration va mener. Toutefois, les sanctions envers ceux qui ne respectent pas les règles ne changeront pas à elles seules la situation de nos agriculteurs. Nous devons veiller à l’application pérenne des lois Égalim. Nous le devons à nos agriculteurs, pour améliorer leur quotidien et faire en sorte que leur travail soit justement reconnu. Monsieur le ministre, comment renforcer l’application des lois Égalim, afin que les négociations commerciales soient équilibrées et que chacun puisse vivre dignement de son travail ? La parole

je partage totalement ce que vous venez de dire sur le revenu des producteurs : c’est, bien évidemment, le combat essentiel. Je l’ai mené comme ministre de l’agriculture pendant trois ans ; je le mène aujourd’hui comme ministre de l’économie et des finances, avec M. le Premier ministre et avec le ministre de l’agriculture, M. Marc Fesneau.

un doublement des contrôles de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur 1 000 contrats, qui concernent 75 des plus gros industriels et les 5 distributeurs. Sur ces 1 000 contrats, 124 ne respectent pas, pour des raisons de calendrier notamment, les dispositions de la loi Égalim. J’ai donc adressé des injonctions à l’ensemble des distributeurs et des industriels qui ne respectent pas les règles ils ont quinze jours pour fournir des explications ou se conformer à la loi, faute de quoi chacun encourra une sanction de 5 millions d’euros par infraction. Croyez moi, nous n’aurons pas la main qui tremble : les sanctions tomberont sur tous les distributeurs et sur tous les industriels qui n’auraient pas respecté strictement et rigoureusement les dispositions de la loi Égalim.

à travailler, à cultiver, à produire en France, sur le territoire français, selon les normes et les réglementations françaises. Encore une fois, nous avons multiplié les contrôles. Les industriels qui s’amusent à mettre des drapeaux tricolores sur des produits qui viennent de l’étranger s’exposent à une sanction qui pourra aller jusqu’à 15 % de leur chiffre d’affaires. Là aussi, les sanctions tomberont et personne ne passera entre les mailles du filet.

Vous devez comprendre que si l’Europe est attaquée, nous ne viendrons jamais pour vous aider et vous soutenir » : ces propos surprenants sont ceux que le président américain Donald Trump a tenus en 2020 à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.

dans quelques mois, si Donald Trump gagne une nouvelle fois les élections, que vaudra encore l’Alliance atlantique ? Au delà des nouvelles adhésions, nous devons absolument nous pencher sur nos capacités. La question des munitions est un enjeu crucial de la guerre de haute intensité. Chaque jour, les Ukrainiens tirent entre 5 000 et 8 000 obus, quand les Russes en tirent exactement le double. Les États européens se sont engagés à soutenir l’effort de guerre ukrainien et à livrer à Kiev 1 million d’obus, c’est à dire, au mieux, six mois de munitions. Nous ne tiendrons pas cet engagement. Nous espérons tout juste pouvoir atteindre la moitié et livrer un peu plus de 500 000 obus avant la fin du mois de mars. Pourquoi ? Non parce que nous n’en produisons pas assez, mais parce que nous continuons collectivement d’en exporter au bénéfice de pays qui en ont bien moins besoin que l’Ukraine.

le chef de l’État s’était engagé à ce que plus personne ne dorme dans la rue. Six ans plus tard, les derniers chiffres de la Fondation Abbé Pierre sont alarmants : ils font état de 330 000 sans abri, dont une proportion croissante de femmes et d’enfants. Il est primordial de comprendre les parcours de vie qui conduisent ces personnes à se retrouver sans domicile fixe. Les raisons peuvent être multiples : perte d’un emploi, difficultés financières, problèmes de santé mentale, ruptures familiales ou encore situations de violence domestique. Ces personnes vulnérables se retrouvent exposées à l’insécurité de la rue et à des conditions de vie très précaires. Les centres d’hébergement sont surpeuplés, les services sociaux sont débordés et les programmes d’aide sont insuffisants. Environ une personne sur deux qui contacte le 115 ne se voit proposer aucune solution d’hébergement. Ayant moi même pris l’initiative d’appeler le 115, en quête d’une solution pour une personne en grande difficulté, je n’ai malheureusement obtenu aucune proposition concrète. Cette situation souligne les lacunes de notre système actuel. Il est du devoir de l’État de trouver des solutions et de mobiliser les ressources nécessaires pour résoudre cette crise sociale grandissante. Nous devons augmenter de manière significative le nombre d’hébergements d’urgence et envisager de réquisitionner les logements vacants, afin de fournir une solution d’urgence et temporaire pour les sans abri et prévenir les situations d’extrême vulnérabilité. Il est primordial de coordonner les actions des différents acteurs impliqués – services sociaux, associations caritatives et collectivités locales –, qui se retrouvent souvent seuls sur le terrain.

que le Gouvernement compte prendre pour remédier à cette situation. Quels sont les projets en cours ou à venir visant à augmenter le nombre de places dans les hébergements d’urgence ? Que comptez vous faire pour renforcer les programmes d’aide aux sans abri et améliorer l’accès aux services sociaux ? La parole est à M. le ministre de la transition

3 milliards d’euros, avec deux types de dispositifs, soit 203 000 places d’urgence – un record – et 114 000 places dans le cadre du dispositif national d’accueil.

au nom du Gouvernement, d’une nouvelle enveloppe de 120 millions d’euros, représentant l’équivalent d’une dizaine de milliers de places. Monsieur le sénateur, je n’ai pas entendu dans votre question

moins. C’est la suite à la fois de décisions qui ont été prises, de textes qui ont été votés et de ce que nous aurons à mettre en œuvre dans les prochaines semaines et les prochains mois.

dix ans après l’appel de l’abbé Pierre que vous évoquiez à l’instant, votre responsabilité est immense et vos réponses ne sont pas à la hauteur. Pas à la hauteur, au moment où le rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre a présenté des chiffres dramatiques : 12 millions de personnes fragilisées par la crise du logement, 4 millions de personnes mal ou non logées, 1 million de personnes dans un habitat indigne et plus de 300 000 personnes sans domicile en France. Pas à la hauteur, au moment où nous n’avons toujours pas de ministre du logement – peut être prochainement ? Pas à la hauteur, enfin, quand M. le Premier ministre, dans son discours de politique générale, aura à peine consacré trois minutes à ce sujet extrêmement important, pour nous proposer finalement – suscitant une consternation partagée par l’ensemble des acteurs concernés, à savoir les maires des plus grandes villes de France, qui vous ont adressé une lettre ouverte, les

tour de passe passe statistique qui cassera le thermomètre de la mixité sociale et dont l’incidence sera quasiment nulle, voire négative, sur la production de logements sociaux dans notre pays. Ma question est simple : comptez vous abandonner cette proposition et enfin mettre en œuvre une politique volontariste et ambitieuse en matière de logement ? Bravo !

entendre, une crise frapperait notre pays, nous serions sur un îlot de déstabilisation et de difficultés, quand dans tous les pays, aujourd’hui, la hausse des taux d’intérêt et l’augmentation des coûts de construction des matériaux ont entraîné une baisse de la production. Et la loi SRU ! En Allemagne, où vos amis sont en responsabilité, la baisse des mises en chantier est comparable à celle de la France. en Chine ou aux États Unis ! Partout ! La loi SRU ! Alors dire que nous aurions un problème français, sincèrement, c’est passer à côté d’une forme de responsabilité.

et avec sincérité, je vais vous exprimer un coup de colère. Un coup de colère, parce que je suis élu d’un département dans lequel le seuil des 100 000 demandeurs de logement Un coup de colère, parce que 12 millions de personnes fragilisées par la crise du logement, ce sont 12 millions de sinistrés. Oui, il s’agit d’une bombe sociale à retardement ! La vérité, c’est que, dès 2017, vos politiques n’ont été qu’un « J’accuse… ! » du logement social, pour libérer de toute contrainte le marché privé baisse des APL dès l’élection du président Macron ; ponction de 1,3 milliard d’euros dans les caisses des bailleurs sociaux ; loi Élan pour obliger à vendre des logements sociaux à la découpe et faire disparaître les petits bailleurs ; loi Kasbarian Bergé pour faciliter les expulsions ; et vous voilà désormais

56 % d’augmentation des loyers dans le parc privé, stop ou encore ? Quelque 2 000 enfants à la rue, stop ou encore ? À quand l’état d’urgence du logement ?

au sein du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, avec Bruno Le Maire, pour expertiser, en particulier, le crédit et le crédit hypothécaire, dispositifs qui, dans des pays voisins, ont permis

de cinq axes : moratoire sur les expulsions, encadrement des prix du foncier, plan pour les primo accédants, relève du niveau de production et réquisition nationale des logements vides. Pour cela, encore faudrait il avoir une ou un ministre du logement. Monsieur le Premier ministre, l’abbé Pierre disait : « Gouverner, c’est d’abord loger son peuple. » Vous êtes le chef du Gouvernement : alors maintenant, vraiment, gouvernez

de la culture, vous avez déclaré la semaine dernière que, pour « préserver » l’audiovisuel public, il faut « rassembler les forces » en un « pôle puissant ». Vos propos rappellent les travaux de l’un de vos prédécesseurs, Franck Riester, qui avait présenté en conseil des ministres un projet de loi autorisant la création d’une holding pour chapeauter l’ensemble des acteurs de l’audiovisuel public. Malheureusement, la crise de la covid 19 a arrêté à l’Assemblée nationale les débats sur ce texte et vos deux prédécesseures,

Il est nécessaire, en effet, de rendre pérennes et définitives ces coopérations, au travers d’une gouvernance commune et d’actions concrètes non seulement dans les fonctions supports, mais aussi dans l’investissement en faveur des nouvelles technologies, en particulier l’intelligence artificielle. Madame la ministre, pour renforcer ces coopérations, il y a trois possibilités. La première, ce sont les contrats d’objectifs et de moyens, tels que l’État les met en œuvre depuis plusieurs années et dont nous savons maintenant qu’ils sont inefficaces. La deuxième, c’est la holding dont je viens de parler.

Vous avez même ajouté, je cite de mémoire : « Ma vie s’est construite avec l’audiovisuel public. » Dès lors, pourquoi ne pas commencer votre action par l’audiovisuel, qui attend une réforme depuis si longtemps ? En effet, la loi de 1986, relative à l’ensemble de l’audiovisuel, est à bout de souffle. L’absence de pluralisme et de réforme du service public menace le consensus national sur la nécessité de lui accorder plus de financements. La réglementation de la production enrichit des fonds d’investissement américains, qui ont mis la main sur de nombreux producteurs français ; et j’en passe… passe… La débureaucratisation promise par M. le Premier ministre a t elle vocation à s’arrêter aux portes de l’audiovisuel français ? La maîtrise de la dépense publique est elle condamnée à ne pas concerner l’audiovisuel public, dernier adepte du « quoi qu’il en coûte » coûte » ? Le principe de libre entreprise est il obligatoirement destiné à ne pas s’appliquer à nos chaînes privées, entravées par des réglementations surabondantes qu’ignorent les plateformes américaines ? En un mot, madame la ministre, formule le Sénat de manière constante depuis 2015 sont elles vouées à être toujours saluées, mais rarement appliquées, par des locataires de la rue de Valois d’autant plus applaudis lors de leur départ que leur bilan aura été minuscule ? La proposition de loi de mon collègue et ami le président Laurent Lafon, dont je fus le rapporteur, adoptée par le Sénat voilà quelques mois, constitue une base solide pour avancer. Madame la ministre, pouvez vous nous préciser vos intentions et, surtout, votre calendrier dans ce domaine ?

Hugonet, pour la réplique. Nous avons entendu, madame la ministre, votre volonté d’ouvrir le débat quant à l’avenir de l’audiovisuel. Il y a urgence, car nous devons notamment nous pencher dès la fin de l’année sur l’avenir de son financement. Autant le dire clairement, les conditions ne sont pas réunies aujourd’hui pour accorder un blanc seing sous la forme d’une modification de la loi organique. Seule une réforme d’envergure garantissant le pluralisme et modifiant la gouvernance pourrait justifier une telle évolution. Vous même avez souligné l’excellence des travaux menés ici, au Sénat, dans ce domaine

De la même façon, vous avez attendu, monsieur le Premier ministre, qu’un autre drame humain se déroule dans mon département, le Puy de Dôme, avec le suicide d’une enfant placée âgée d’à peine 15 ans, pour prendre enfin les décrets d’application d’une loi votée voilà deux ans.

nous, demain, un ministre de l’enfance de la protection de l’enfance, un ministre doté des moyens financiers pour engager, enfin, ce plan Marshall de la protection de l’enfance qui est plus qu’urgent, avec tous les acteurs concernés, et pour « désinvisibiliser » ces 350 000 enfants placés et les professionnels qui les accompagnent sans relâche ?

Rien lors de votre déclaration de politique générale, monsieur le Premier ministre. Rien pour les 350 000 enfants placés, dont 10 000 bébés, certains atteints du syndrome de l’hospitalisme. Rien pour la santé mentale de ces enfants, qui perdraient vingt ans d’espérance de vie et font trente sept fois plus de dépressions et de tentatives de suicide. Rien sur la reconnaissance de l’utilité sociale des professions de la protection de l’enfance. Rien pour les départements en première ligne et qui font face à un resserrement de leurs finances. Le propre de la puissance est de protéger, écrivait pourtant Blaise Pascal. Votre gouvernement semble toujours plus prompt à réprimer qu’à protéger. J’en veux pour preuve que les décrets d’application relatifs au code de la justice pénale des mineurs ont, eux, été pris en trois mois, quand il a fallu attendre deux ans

La parole est à M. Georges Naturel, pour le groupe Les Républicains.

Monsieur le ministre, la filière du nickel en Nouvelle Calédonie traverse actuellement une crise d’une rare gravité. Les trois usines métallurgiques de Koniambo Nickel SAS (KNS), de la Société Le Nickel (SLN) et du Sud connaissent depuis plusieurs mois des difficultés majeures et sont au bord du dépôt de bilan. Plusieurs milliers d’emplois directs et indirects sont en cause et de très nombreuses familles calédoniennes vivent dans l’angoisse de lendemains particulièrement difficiles. La fermeture de l’usine de KNS, aujourd’hui la plus menacée avec environ 1 300 emplois directs,

Monsieur le ministre, pouvez vous nous indiquer précisément quel est, à ce jour, l’état des négociations de ce pacte Nickel ? Pour chacune des usines, avez vous obtenu de la part des actionnaires Eramet pour la SLN, Glencore pour KNS et Trafigura pour l’usine du Sud – les engagements que vous demandez ? Avez vous obtenu l’accord de tous les élus calédoniens pour que la ressource minière soit mieux valorisée ? Quand allez vous annoncer, pour chacune des usines, le montant et la date du déblocage des prêts relais de l’État ? Enfin, quand allez vous annoncer les modalités et le calendrier du soutien de l’État pour moderniser la production d’électricité et réduire son coût ?

je partage totalement votre diagnostic sur l’état de la filière du nickel en Nouvelle Calédonie, confrontée à la fois à une concurrence nouvelle de la part de l’Indonésie, de la Corée du Sud, de la Chine, qui produisent à des coûts bien inférieurs, et à un effondrement du cours du nickel. mettent les trois usines, celle du Sud, celle de Nouméa et celle du Nord, en grande difficulté. Je me suis rendu sur place avec le ministre de l’intérieur et des outre mer, Gérald Darmanin, voilà quelques semaines, pour faire le point avec l’ensemble des acteurs, les élus et les industriels. J’ai dit à quel point je croyais dans l’avenir économique de la filière du nickel en Nouvelle Calédonie.

Deuxième condition : il convient que l’État s’engage sur la rénovation des réseaux électriques. Le Président de la République a pris de tels engagements et je suis chargé de les mettre en œuvre. Nous mobiliserons les investissements nécessaires pour moderniser le réseau énergétique calédonien. Troisième condition, essentielle

45 millions d’euros d’aide immédiate, 65 millions d’euros de soutien sous une autre forme financière, soit près de 200 millions d’euros de soutien pour une seule usine.

que des grands groupes producteurs d’eaux minérales utilisaient en fait des traitements qui n’étaient pas autorisés auparavant pour les eaux de source.

Lorsque les informations nous ont été relayées, les agences régionales de santé ont saisi le procureur de la République pour risque de manquement à la réglementation et tromperie du consommateur. Une eau minérale doit respecter

Une enquête judiciaire a été ouverte et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes apporte son soutien à cette enquête pour examiner si, oui ou non – je n’ai évidemment pas la réponse

Cette loi affecte, entre autres, les animaleries, les cirques, les parcs zoologiques, les parcs aquatiques. Les professionnels concernés sont talentueux, passionnés, soucieux du bien être des animaux qu’ils hébergent, soignent et étudient. Depuis 2021, les textes réglementaires concernant les parcs aquatiques accueillant les mammifères marins ne sont toujours pas signés. Promenés de secrétaire d’État en secrétaire d’État à la faveur des remaniements ministériels, ces parcs n’ont pas de ligne claire sur le cadre applicable à leurs activités et n’ont, de ce fait, aucune assurance que celles ci soient pérennes. Ce n’est pas l’esprit de la loi qui a été votée.

Pouvez vous nous dire quand, enfin, les arrêtés concernant les conditions d’hébergement, les contours des programmes scientifiques et les démonstrations au public des résultats des recherches seront signés ?

qui sont notre patrimoine. Ils font la fierté de la France. La Haute Assemblée veillera à ce que la France reste la France ! La parole est à M. Hervé Gillé, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

voilà les faits qui sont reprochés au Gouvernement à la suite des révélations de Radio France et du journal à la fin du mois de janvier. Cette enquête nous informe qu’un rendez vous s’est tenu en 2021 entre Nestlé Waters et le cabinet de Mme Pannier Runacher, alors ministre déléguée chargée de l’industrie. À la

L’enquête judiciaire est ouverte. La justice a été saisie par les ARS au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes va apporter son expertise pour déterminer la conformité ou non de ce qui a été décidé par les industriels, et la justice rendra sa décision dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Laissons la justice mener son enquête jusqu’au bout : elle est la seule à même, désormais, à pouvoir apporter des réponses à vos questions.

en quelque sorte, les conditions d’une société de défiance et de suspicion. Pis, ce type de comportement peut alimenter les théories du complot. Si vous souhaitez clarifier la situation, vous ne pourrez que soutenir la création d’une commission d’enquête parlementaire sur le sujet. Nous jugerons donc sur les actes.

Ma question s’adresse au ministre de l’intérieur et des outre mer. Monsieur le ministre, notre groupe est profondément préoccupé par la situation de chaos dans laquelle vit Mayotte et sur laquelle, du reste, nos collègues mahorais vous alertent régulièrement. La crise La crise de l’eau récemment très médiatisée s’est en réalité ajoutée à l’insécurité, à la pauvreté, à l’insalubrité, à l’immigration galopante, à une crise économique et sociale profonde, aux difficultés liées aux infrastructures sous dimensionnées. La population, excédée, paralyse une nouvelle fois Mayotte pour protester contre l’insécurité. Cette situation insurrectionnelle n’est pas plus acceptable à Mayotte qu’ailleurs dans notre République. Rétablir durablement la sécurité et l’autorité de l’État doit être la première des priorités. L’immigration incontrôlée est à l’origine de la pression démographique : il naît l’équivalent d’une classe par jour à la maternité. Il faut certes durcir les règles d’immigration et d’acquisition de la nationalité en vigueur à Mayotte et tarir ainsi la principale difficulté mais on ne peut plus se contenter de mesures d’urgence, qui permettent seulement d’apaiser les tensions pour un temps. On voit bien que Mayotte a besoin d’une vision pour adapter efficacement et structurellement l’action de l’État et des collectivités locales à sa réalité. Sans moyens, le droit ne peut s’appliquer efficacement. Un projet de loi pour un développement accéléré de Mayotte avait été annoncé en 2021. Nous sommes en 2024 et le désespoir s’empare de la population. Eu égard au caractère multidimensionnel de la crise, monsieur le ministre, êtes vous en mesure de nous annoncer un plan ou une loi de programmation pour Mayotte ?

appartenant au conseil départemental et, pour la première fois, de rapatriement dans l’Hexagone de personnes reconnues comme réfugiées par le droit d’asile français. Par ailleurs, le Premier ministre a annoncé dans son discours de politique générale

Mayotte, comme l’ensemble des outre mer, a besoin d’un projet ambitieux, car la situation est aussi le résultat d’une gestion par à coups et à trop court terme. Je suis persuadée que l’on paie plus cher à long terme et à tout point de vue – ce que l’on repousse d’année en année. À Mayotte, le Gouvernement doit donc s’attaquer aux causes profondes, au premier rang desquelles l’immigration.

Aucun des 283 passagers n’a survécu. Depuis le 1 février 2024, Pékin met en danger la sécurité aérienne dans le détroit de Taïwan. Un vol Air France passe par ce couloir aérien. L’administration de l’aviation civile chinoise a décidé, unilatéralement, d’une modification de ses itinéraires de vol dans le couloir aérien M503, qui viennent désormais frôler la frontière aérienne officieuse entre Taïwan et la Chine. L’objectif de Pékin est clair : harceler les défenses aériennes de Taïwan et se servir du passage d’avions civils pour camoufler des manœuvres militaires. Taïwan condamne cette décision et pointe les conséquences néfastes en termes de sécurité des passagers internationaux, dont nos ressortissants, en provenance et à destination de Shanghai. La révocation de l’accord aérien conclu en 2015 entre les deux rives du détroit de Taïwan constitue un coup de force et porte atteinte au.

que fera la France pour amener la Chine à revenir à l’accord aérien conclu avec Taïwan en 2015 et sécuriser ainsi nos ressortissants ? La parole

que la France porte d’ailleurs à un haut niveau auprès des autorités chinoises, en les encourageant à privilégier le dialogue et à éviter toute escalade. La France est attachée à la paix et à la sécurité de la région. Cette position se traduit par le passage régulier de notre marine nationale dans les eaux internationales du détroit.

Brigitte Devésa, pour la réplique. Nul n’est dupe ici : la Chine, irritée par le résultat de la présidentielle à Taïwan, cherche désormais à instrumentaliser l’aviation civile pour des considérations politiques et militaires.

La séance est suspendue.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

Madame la présidente, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, vous le savez, la France paie chaque année un lourd tribut au tabagisme. C’est la première cause de mortalité évitable avec 75 000 décès par an, soit 200 morts par jour. Selon l’Institut Curie, si tous les moins de 20 ans arrêtaient de fumer demain, la mortalité par cancer diminuerait de 40 % dans les cinquante

dans notre société. Nous portons depuis plusieurs années une attention particulière à l’entrée des jeunes dans le tabagisme. Nous allons dans le bon sens : chez les jeunes de 17 ans, la prévalence du tabagisme quotidien a baissé significativement entre 2017 et 2022 de 25,1 % à 15,6 %. Cependant, les jeunes générations demeurent la cible prioritaire de l’industrie du tabac. L’addiction nicotinique est d’autant plus forte qu’elle est initiée précocement. En France, l’âge moyen de la première cigarette se situe aujourd’hui aux alentours de 14 ans. Il est particulièrement important d’agir résolument face aux nouvelles tendances, dont font partie les produits de vapotage. Ils posent des risques importants d’entrée dans la dépendance à la nicotine. Je veux donc saluer ce texte, qui vise à l’interdiction des dispositifs électroniques de vapotage à usage unique. Le marketing de ces produits est conçu pour attirer les jeunes, avec ses couleurs, ses parfums ses parfums et ses prix bas. Nous voyons des dispositifs arriver sur le marché dont le contenu équivaut à dix huit paquets de cigarettes. C’est un danger sanitaire pour les plus jeunes. Chez les 13 16 ans, on estime qu’un jeune sur dix a déjà essayé la « La puff n’est pas un dispositif de sevrage. Son taux de nicotine pouvant aller jusqu’à 20 milligrammes par millilitre ouvre la voie à une forte dépendance. Elle apprend aussi le geste de fumer. Tous ces éléments facilitent l’effet passerelle vers le tabagisme. Nous allons mettre en place une veille sur tous les nouveaux produits du tabac et du vapotage. Je pense aux sachets de nicotine, arrivés récemment. Ce combat nécessite de l’engagement

Un territoire de la République en a déjà interdit l’importation : la Nouvelle Calédonie. Nos voisins belges, allemands ou irlandais sont en train de mettre en place des interdictions similaires à celle que nous examinons aujourd’hui. C’est une politique de prévention indispensable face aux enjeux que j’évoquais. Le 22 juin 1976, dans cet hémicycle, Simone Veil défendait le projet de loi de lutte contre le tabagisme, en évoquant l’importance de combler notre « retard sensible en ce qui concerne la prévention et, tout particulièrement, l’information et l’éducation sanitaires ». Elle ajoutait que « limiter la politique de santé à la seule médecine de soins – si essentiel que soit son rôle – en s’abstenant de remédier, lorsque c’est possible, aux causes mêmes des maladies, serait à la fois illogique et injustifié aussi bien sur le plan humain que du point de vue économique Tout était dit, mesdames, messieurs les sénateurs. Ce combat pour la prévention, nous le poursuivons aujourd’hui. En matière de prévention du tabac, nous avons tout un arsenal de mesures, détaillé dans le plan national de novembre 2023. Pour protéger les jeunes du tabagisme, nous avons pris des mesures fortes de rendre le tabac moins accessible, moins attractif et moins abordable. Pour accompagner les fumeurs, en particulier les plus vulnérables, nous renforçons les mesures de repérage, d’information et d’accès aux traitements de substitution. Pour protéger notre environnement, nous instaurons de nouveaux espaces extérieurs à usage collectif sans tabac. Pour transformer les métiers du tabac et lutter contre les trafics, nous soutenons les buralistes face aux évolutions de leur métier et nous renforçons notre lutte contre le marché parallèle. Enfin, pour améliorer la connaissance sur les dangers liés au tabac et les interventions pertinentes, nous renforçons activement le domaine de la recherche. Le Président de la République l’avait annoncé lors de la journée mondiale contre le cancer de 2021 : nous visons une génération sans tabac dans les années 2030. Soyez assurés que je mettrai toute mon énergie et toute celle de mon ministère au service de cet objectif. C’est un défi de santé publique, mais plus largement un défi sociétal. Nous devons

La proposition de loi qu’il nous revient d’examiner a été votée à l’Assemblée nationale à l’unanimité le 4 décembre dernier. Composée d’un article unique, elle n’en est pas moins porteuse d’enjeux sensibles et mérite toute notre attention. notre attention. La France est le troisième marché mondial de la cigarette électronique : il représente un chiffre d’affaires de près d’un milliard d’euros et compte plus de 3 millions de vapoteurs. Les cigarettes électroniques jetables, ou puffs, représentent un nouveau segment de ce vaste marché. Elles connaissent en France un succès grandissant depuis 2021.

Sous une apparence inoffensive, les puffs dissimulent pourtant un produit loin d’être anodin et des stratégies commerciales très offensives. Avec ces dispositifs, les industriels cherchent non pas à convertir des fumeurs traditionnels à un autre produit, mais bien à capter de nouveaux consommateurs de nicotine. Nous ne devons donc pas nous laisser berner par le discours fallacieux de la réduction des risques qu’ils ont élaboré : 80 % des puffs vendues en France contiennent de la nicotine. Dans la tranche des 13 16 ans, 15 % déclarent avoir déjà utilisé une puff et 47 % d’entre eux disent avoir commencé leur initiation à la nicotine avec ce produit. La nicotine est une drogue dure et une drogue triste. Dure, parce qu’elle induit une dépendance très forte et une dégradation de la santé mentale de ses usagers. Triste, parce qu’elle n’a pas d’effet euphorisant, bien au contraire. Les jeunes, dont le développement cérébral n’est pas encore à maturité, sont particulièrement vulnérables à ces effets. Contenue sous forme de sels dans les puffs, l’inhalation de la nicotine se trouve facilitée, ce qui peut conduire à en absorber des quantités plus importantes qu’avec le tabac. De plus, les aldéhydes, ces substances néo chauffées issues de la combustion partielle du liquide, sont probablement toxiques et cancérigènes, mais nous manquons de recul à ce jour pour consolider les données scientifiques existantes. Les puffs s’achètent partout. Peu onéreuses, elles sont un produit accessible aux adolescents. Les modèles les plus récents, qui se retrouvent aussi sur le marché français, ne respectent pas tous les normes en vigueur, qu’il s’agisse du format du réservoir, limité à 2 millilitres, ou du taux maximal de nicotine, fixé à 20 milligrammes par millilitre. Nos législations nationales sont mises à l’épreuve, car elles peinent à suivre les évolutions du marché. C’est pourquoi il nous incombe d’être vigilants pour proposer un texte suffisamment agile et englobant. Vous l’aurez noté, l’interdiction porte à la fois sur la fabrication, la vente et la distribution ou l’offre à titre gratuit. Si la question d’une éventuelle interdiction

D’ailleurs, dès lors que la fabrication et la vente ou la cession de ces produits sont interdites, l’intérêt de les importer ne pourrait recouvrir que des hypothèses très limitées, voire théoriques. Je rappelle que les puffs sont aujourd’hui fabriquées en Chine et qu’il n’existe pas de filière de production en France. On peut regretter que l’interdiction de vente aux mineurs des produits du tabac et du vapotage ne soit que très imparfaitement respectée. Pourtant, cette proposition de loi n’est pas un aveu d’échec et constitue une réelle avancée. En effet, l’interdiction générale des dispositifs électroniques de vapotage à usage unique sera plus aisée à contrôler qu’une interdiction circonscrite aux seuls mineurs l’amende de 100 000 euros qui sanctionne le non respect de l’interdiction est véritablement dissuasive. Il n’en demeure pas moins indispensable d’accompagner la mise en œuvre du texte de moyens de contrôle appropriés, pour garantir son effectivité. Ces moyens apparaissent notoirement insuffisants aujourd’hui. La vente sur les réseaux sociaux et l’ubérisation du commerce ont rendu tout produit aisément accessible. En tant que membre de la commission d’enquête sur le narcotrafic, je suis particulièrement sensibilisé à ces questions et soucieux de réfléchir aux moyens les plus efficaces pour empêcher les contournements de la loi. À ce titre, je crois que nous pourrions envisager une mesure de contrôle de la majorité lors de l’achat en ligne des produits du tabac ou du vapotage, même si le sujet est complexe, j’en ai conscience.

Le volume a donc été multiplié par quatre en une année. Cette accumulation de nouveaux déchets, qui ne répond à aucun besoin essentiel, doit nous interpeller. Ces cigarettes électroniques jetables sont composées d’une batterie de lithium non amovible. Nous épuisons donc consciemment des ressources naturelles sensibles pour créer des produits nocifs, à la durée de vie excessivement courte. L’indécence de ce modèle doit nous amener Pis : ces déchets, qui s’amoncellent, sont en pratique presque impossibles à recycler, principalement du fait de l’inamovibilité de leur batterie. Quant au lithium, il est à la source de départs d’incendies réguliers dans les centres de tri et de traitement des déchets et expose les biens et les personnes à des risques importants. Ce risque se trouve donc démultiplié avec les puffs. Pour finir, j’évoquerai l’enjeu que représente cette proposition de loi au regard de l’Union européenne. Cette interdiction des dispositifs de vapotage à usage unique ne pourra entrer en vigueur que si la Commission européenne l’approuve. En effet, en application du principe de libre circulation des marchandises, un État membre de l’Union n’est fondé à interdire un produit conforme à la réglementation européenne

envisagent une interdiction similaire en Europe. Il est donc essentiel que la France affirme une volonté politique forte en faveur de l’interdiction des puffs. Au moment où des travaux sont engagés pour actualiser la directive européenne sur les produits du tabac, sa voix doit porter pour être entendue. Vous l’avez compris, mes chers collègues, l’article unique de cette proposition de loi est lourd d’enjeux. Les auditions menées et l’instruction du texte ont renforcé ma conviction et ma détermination à vous convaincre de l’intérêt d’adopter cette proposition de loi. Pour finir, à ceux qui invoqueraient un risque de report des usagers de la cigarette électronique jetable vers le tabac, je souhaite répondre qu’il est de notre responsabilité – vous l’avez rappelé, madame la ministre – de poursuivre et d’accentuer nos efforts

Si nous pouvons nous satisfaire de cette amélioration, nous devons rester vigilants et agiles. L’industrie du tabac ne cesse, en effet, de multiplier les innovations pour attirer les plus jeunes de nos concitoyens dans les filets du tabagisme. L’objet du débat qui s’ouvre en est un exemple frappant. Les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique, dits puffs, se sont imposés dans notre société à une vitesse grand V, en particulier chez nos jeunes jeunes : 15 % des adolescents de 13 à 16 ans auraient déjà utilisé une puff, et 47 % de ces jeunes usagers déclarent avoir commencé leur initiation à la nicotine avec ce produit. Par ailleurs, en novembre dernier, les cigarettes électroniques jetables représentaient près de 30 % des références notifiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, contre moins de 4 % à Il nous faut le dire haut et fort : oui, la puff est en train de devenir un fléau pour nos jeunes ! Elle explique l’importance de la proposition de loi que nous examinons. En interdisant la fabrication, la vente, la distribution et l’offre gratuite des dispositifs électroniques de vapotage à usage unique en France, nous répondrons à une double préoccupation, à la fois sanitaire et environnementale.

Diverses études démontrent le caractère fortement addictif de la nicotine et l’associent à des troubles anxiodépressifs et à une dégradation de la santé mentale chez ses usagers.

Cela ouvre la voie à une forte dépendance et crée une accoutumance au geste de fumer, ce qui facilite l’effet passerelle vers le tabagisme. La puff constitue aussi un modèle commercial décomplexé et agressif, qui cherche à recruter de nouveaux consommateurs chez les adolescents. Elle est très accessible, étant à la fois facile à utiliser et peu onéreuse, avec un prix variant entre 8 euros et 12 euros pour 600 à 2 000 bouffées. Colorées et ludiques, les puffs ont des saveurs sucrées et fruitées, qui ciblent clairement les jeunes. Les réseaux sociaux, notamment TikTok et Instagram, en font une promotion active, malgré l’interdiction de toute publicité en faveur des produits du vapotage. Deuxièmement, la puff est à contre courant des enjeux de transition écologique. La composition des puffs, fabriquées avec des plastiques et métaux lourds, en fait des déchets particulièrement polluants. Bien qu’ils soient le plus souvent jetés avec les ordures ménagères, ils constituent des équipements électriques et électroniques, qui relèvent d’une filière spécifique de

que les produits disposent de batteries facilement amovibles. Par ailleurs, le traitement du lithium dans les centres de tri et de recyclage comporte des risques d’incendie importants, qui menacent la sécurité des travailleurs : en moyenne, un centre de tri est détruit chaque année en France ! Nous devons aussi constater que la législation en vigueur est plutôt un échec. Je rappelle que la publicité sur les produits du vapotage, qu’ils soient jetables et qu’elle est assortie d’une interdiction de vente aux mineurs et d’une interdiction de vapoter dans certains espaces, dont les établissements scolaires. Pourtant, les enquêtes démontrent que l’interdiction de vente aux mineurs est régulièrement enfreinte. Plus d’un quart des adolescents mineurs estiment qu’il est facile d’acheter et de se procurer des puffs. Cette difficulté manifeste à opérer des contrôles et à réaliser des constats de flagrance pour sanctionner le non respect de la loi pose,, la question des moyens et du caractère dissuasif des sanctions. Il est donc essentiel de se doter d’un cadre législatif englobant et agile face à l’émergence de nouveaux usages, dont la puff fait partie. Tel sera le cas si nous adoptons cette proposition de loi, notamment grâce aux avancées obtenues en commission sur la définition du dispositif électronique jetable à usage unique ou encore sur la sanction du non respect de l’interdiction de fabriquer des puffs. mes chers collègues, le groupe RDPI se positionne clairement en faveur de ce texte. Néanmoins, la seule interdiction des dispositifs électroniques de vapotage à usage unique ne résoudra pas tous les problèmes liés au tabagisme en France. Le précédent ministre de la santé et de la prévention, Aurélien Rousseau, avait annoncé un double objectif dans le cadre du programme national de lutte contre le tabac (PNLT) : faire apparaître une génération sans tabac d’ici à 2032 et accompagner les fumeurs dans l’arrêt du tabac. Ce sujet de société nous concernant tous, il est essentiel de mener un travail collectif, pour pour avancer au delà de nos clivages. Nous devons aussi mieux anticiper l’avènement de nouveaux produits, comme le tabac à chauffer, le tabac à mâcher ou les sachets de nicotine. Renforçons notre action à destination des fumeurs pour les aider à arrêter le tabac et mieux les accompagner, car, ne l’oublions pas, ce sont encore 200 Français qui meurent chaque jour à cause du tabac. Les mots de Claude Évin sont plus que jamais d’actualité : la lutte contre le tabagisme « a toujours eu eu dans nos institutions une valeur symbolique. Sans doute parce qu’il s’agit de légiférer sur des comportements, des activités et des habitudes de vie qui conduisent à la mort ou à la souffrance physique et psychologique. » À cet égard, si la présente

Ce texte est transpartisan, puisqu’il a recueilli, à l’Assemblée nationale, la signature de députés venant de huit groupes politiques. À notre Haute Assemblée, maintenant, de se prononcer ! Je veux, pour commencer, saluer la qualité du travail du rapporteur de notre commission des affaires sociales, M. Khalifé.

ne contiennent pas de tabac, mais peuvent renfermer de la nicotine, substance au double effet psychotrope et addictif. Bien évidemment, cette proposition de loi ne s’attaque pas aux produits de vapotage rechargeables qui servent à sortir de la consommation de tabac ni aux nouvelles formes de délivrance nicotinique. Il est urgent d’interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique, car ce sont les adolescents qui sont visés par de tels produits, alors même que leur vente est interdite aux mineurs. Format minimaliste, facilement dissimulable aux parents, multitude de goûts disponibles : le gabarit des puffs et leur design ludique plaisent beaucoup, avec un très fort risque d’addiction.

afin d’attirer les jeunes et, ainsi, de compenser la diminution de la consommation de tabac chez les jeunes générations. Selon Alliance contre le tabac, 28 % des adolescents utilisant la puff ont commencé leur initiation à la nicotine à travers ce produit, et 17 % d’entre eux se sont ensuite tournés vers une autre forme de produit de la nicotine ou du tabac. Il est urgent d’agir, car 15 % des jeunes âgés de 13 à 16 ans ont déjà utilisé une puff. souligne M. Frédéric Le Guillou, pneumologue et président de l’association Santé respiratoire France, les puffs sont « une porte d’entrée dans l’addiction à la nicotine dans un premier temps, et dans l’addiction au tabac dans un second temps. La gestuelle est également responsable d’une dépendance comportementale. » Il est d’autant plus urgent d’agir que les industriels du tabac rivalisent d’inventivité pour tenter de préserver leurs profits mortifères. J’insiste sur le terrible chiffre de 200 morts par jour en France à cause du tabac dernière invention en date est la 9K, une nouvelle puff ultrapuissante qui contient 9 000 bouffées, ce qui équivaut à 18 paquets de cigarettes à 2 % de nicotine ; le packaging est là encore attrayant pour les jeunes, avec des vapoteuses colorées et parfois clignotantes. La démarche des industriels du tabac est extrêmement perverse, comme le souligne l’Académie nationale de médecine : les puffs sont des pièges particulièrement sournois pour les enfants et les adolescents.

boissons contenant de l’alcool masqué par un mélange de jus de fruits très sucré. Quel cynisme, là aussi, pour tenter d’augmenter encore et toujours les profits ! Les buralistes n’ont pas le droit de vendre des puffs 9K, encore moins à des mineurs. Je tiens, d’ailleurs, à souligner la position très responsable des buralistes, qui sont favorables à l’interdiction des puffs. Ces professionnels jouent un rôle primordial dans le maintien du lien social, en particulier dans nos bourgs et nos villages.

et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, texte dont les députés socialistes sont à l’origine et qui a interdit la promotion de tels dispositifs sur les réseaux sociaux. les réseaux sociaux. Si les puffs ont un coût moral, affectif et humain, elles ont aussi un coût potentiel pour notre sécurité sociale, puisqu’elles peuvent être à l’origine de maladies, dont des cancers. Rappelons que le tabagisme est la première cause de mortalité évitable en France : il a été responsable de la mort de 75 000 personnes en 2015. Les puffs ont également un coût environnemental très fort : le plastique et le lithium qui les composent sont très consommateurs de pétrole et d’eau, extraits à l’autre bout du monde, bien souvent en Chine. Les puffs sont donc ultratoxiques pour l’environnement. Jetables, elles sont en plastique et contiennent une batterie au lithium non recyclable. Les cigarettes électroniques à usage unique sont facilement inflammables et constituent des déchets complexes, mal collectés, mal recyclés, présents dans les sols, les nappes phréatiques et les océans. C’est un véritable contresens écologique. L’usage et la durée de vie de ces produits vont à l’encontre des actions et des mesures pour lutter contre le gaspillage, la surconsommation et le réchauffement climatique. le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain du Sénat est tout à fait favorable à cette proposition de loi. Nous voterons pour interdire la fabrication, la vente, la distribution et l’offre à titre gratuit des dispositifs électroniques à usage unique, en y incluant les dispositifs rechargeables susceptibles d’être réutilisés jusqu’à épuisement du liquide prérempli dans le réservoir au moment de l’achat.

L’interdiction des puffs est soutenue par une multitude d’acteurs : citoyens, scientifiques, associations, entreprises de vapotage et buralistes. Il faut faire cesser ces scandales sanitaires et environnementaux que sont les puffs. de loi définitivement adoptée par le Parlement, il appartiendra au Gouvernement, madame la ministre, de notifier à la Commission européenne la mesure d’interdiction des dispositifs électroniques de vapotage à usage unique. Cette notification est nécessaire, puisque les biens et les services circulent librement dans le marché commun. Une interdiction est possible au niveau européen, sous réserve qu’elle réponde à des motifs relatifs à la situation spécifique de l’État concerné et à condition d’être justifiée

La proposition de loi que nous nous apprêtons à examiner vise à interdire les dispositifs électroniques de vapotage jetables ou à usage unique, dits puffs. L’interdiction visée par ce texte s’appliquera à la fabrication, la vente, la distribution et l’offre à titre gratuit de ces dispositifs. En premier lieu, je tiens à souligner que les puffs sont une aberration environnementale, du fait de la nature même du dispositif : ces cigarettes électroniques jetables sont composées principalement de matières plastiques et d’une batterie non amovible, le plus souvent au lithium. Les puffs usagées sont donc, par nature, des « déchets d’équipements électriques et électroniques » (DEEE), qui nécessitent un recyclage spécifique. Or une part importante de ces dispositifs de vapotage jetables ou à usage unique échappe à la filière de retraitement, alors que ces déchets représentent un danger pour l’environnement. Qui plus est, du fait de la petite taille de ces équipements et de leur batterie incorporée, il est impossible de procéder à leur dépollution, sauf à y consacrer des moyens très importants. Quant au lithium, il est à l’origine de départs d’incendies réguliers dans les centres de tri et de traitement des déchets, mettant ainsi en péril la santé des travailleurs. Ensuite, il est évident que ces dispositifs constituent des risques majeurs en matière de santé publique, notamment pour la santé des jeunes. Les puffs sont plébiscitées chez les adolescents. L’usage quotidien de la cigarette électronique a triplé entre 2017 et 2022 chez les jeunes de 17 ans, pour s’établir à 6,2 %. En 2022, l’Alliance contre le tabac indiquait que 13 % des adolescents âgés de 13 à 16 ans avaient déjà utilisé une puff et que, pour 28 % d’entre eux, cela correspondait à leur première consommation de nicotine. L’apparition des cigarettes électroniques jetables fait également évoluer les représentations associées à la cigarette et au tabac chez les jeunes. Vantées pour leur simplicité d’utilisation par les professionnels du secteur, les puffs sont rapidement devenues populaires auprès des enfants et des adolescents, grâce à leurs prix compétitifs, leurs emballages attractifs et leurs saveurs sucrées et fruitées. (Opecst) sur les nouveaux produits du tabac ou à base de nicotine identifie une corrélation entre l’utilisation de cigarettes électroniques et l’entrée dans le tabagisme, en raison du phénomène de dépendance au geste de vapotage, qui peut représenter un nouveau mode d’entrée dans l’addiction tabagique, mais aussi du fait de l’usage de puffs contenant de la nicotine. Ainsi, 47 % des jeunes se sont initiés à la nicotine par la puff, soit près d’un sur deux. Enfin, l’interdiction de la vente aux mineurs est très peu respectée. Selon l’Académie nationale de médecine, ces dispositifs constituent « un piège particulièrement sournois pour les enfants et les adolescents ». Or le tabagisme est le premier facteur de risque évitable de cancer. Chaque année, 68 000 nouveaux cas de cancer, entraînant 40 000 décès, concerne la toxicité des puffs, la plupart des experts s’accordent pour affirmer que les émissions produites par les cigarettes électroniques sont moins nocives que la fumée du tabac. Toutefois, cette moindre nocivité n’est pas synonyme d’absence de toute dangerosité, car le mode d’exposition complexifie l’évaluation des risques. En effet, de nombreux arômes sont considérés comme sûrs lorsqu’ils sont ingérés par voie orale, mais leur innocuité n’est pas nécessairement établie après chauffage et inhalation. L’interdiction des puffs est donc un impératif de santé publique. Toutefois, en application du principe de libre circulation des marchandises, cette interdiction ne pourra entrer en vigueur que si la Commission européenne l’approuve. La position de la France est scrutée par les institutions européennes, mais aussi par des pays qui envisagent la même interdiction – je pense notamment à l’Allemagne et à l’Irlande. je tiens à saluer le travail du rapporteur, qui a consolidé le texte en précisant la définition de ce qu’est un dispositif de vapotage jetable ou à usage unique, afin de circonscrire l’interdiction qui sera examinée par la Commission européenne.

colorés, aromatisés à la fraise, à la pastèque ou encore à la mangue, on pourrait très facilement les confondre avec un paquet de bonbons : les emballages des cigarettes électroniques à usage unique, dites puffs, ne laissent aucun doute sur leur cible marketing : les jeunes. Cependant, un chiffre doit nous réjouir : la diminution de la consommation de tabac chez ces derniers. En effet, en 2022, moins d’un jeune sur deux déclarait avoir déjà fumé, contre près de 60 % en 2017. Aujourd’hui, 16 % des jeunes de 17 ans fument tous les jours, soit deux fois moins qu’il y a dix ans. Quelles que soient les origines de la diminution de la consommation efficacité des campagnes de prévention, augmentation du prix du paquet, loi Évin, pandémie de covid 19… –, nous ne pouvons que nous féliciter de cette baisse. La nocivité du tabagisme est un fait indiscutable : celui ci est la première cause évitable de mortalité prématurée. En France, quelque 45 000 personnes décèdent chaque année d’un cancer lié au tabac. Cette baisse de la consommation a parallèlement ouvert la porte à la cigarette électronique, qui s’est développée à grande vitesse : le vapotage a triplé en cinq ans. Chez les jeunes, depuis 2021, c’est précisément le recours à la cigarette électronique à usage unique qui rencontre un vrai succès. Le packaging est, paraît il, séduisant… Surtout, la vente à l’unité permet un prix bien inférieur à celui d’un paquet de cigarettes, qui, aujourd’hui, coûte environ 11 euros et offre l’équivalent de 300 bouffées. La puff est, quant à elle, accessible à partir de 7 euros pour 800 bouffées, soit plus de deux fois et demie de bouffées supplémentaires, pour un prix inférieur d’environ 36 %. Selon les professionnels, et contrairement à ce que l’on croit, la cigarette électronique, censée ne dégager ni goudron ni monoxyde de carbone, est loin d’être inoffensive. Elle peut contenir de la nicotine et d’autres substances toxiques, tel l’acide benzoïque, dont on ne connaît pas encore les effets sur le long terme. Et le vapoteur d’une puff avec nicotine en absorbe autant que le fumeur de cigarettes classiques… mondiale de la santé (OMS) comme un produit nocif et addictif. Cependant, la littérature scientifique n’est pas unanime sur le niveau de toxicité de la cigarette électronique. Hélas, aucune étude scientifique ne permet, à ce jour, d’affirmer qu’elle est moins dangereuse que la cigarette classique. Je souhaite en profiter pour remercier notre rapporteur. Monsieur Khalifé, vous nous avez aussi alertés sur le fait que les puffs ne s’adressaient pas seulement à des fumeurs voulant réduire leur consommation.

Si la cigarette électronique a des effets néfastes sur la santé, sa version jetable est, quant à elle, pour reprendre l’expression de l’auteur de la proposition de loi, une « véritable aberration puffs nuisent gravement à l’environnement. On sait déjà que la durée de vie d’un mégot est de douze ans. Alors que 23,5 milliards de mégots sont jetés dans l’espace public chaque année en France, coût, pour les collectivités locales, de 100 millions d’euros par an. Les puffs, quant à elles, contiennent du plastique, mais aussi des métaux lourds, comme le lithium, le chrome, le nickel, le mercure, le cobalt, le fer, l’aluminium, le cuivre, le zinc ou encore le plomb – rien que cela D’après les spécialistes, il est quasiment impossible de les recycler, en raison de techniques de fabrication dont je vous épargne les détails. Interdire un produit qui nuit autant à la santé de nos enfants qu’à celle de l’environnement est une évidence.

Le 28 novembre dernier, Aurélien Rousseau, alors ministre de la santé et de la prévention, présentait devant des élus et des journalistes les principaux axes du nouveau programme national de lutte contre le tabac pour la période 2023 2027. Il y était précisé que les résultats du précédent PNLT étaient concluants, puisque 2 millions de fumeurs quotidiens en 2018 ont cessé leur consommation en 2022. Ces chiffres, très encourageants, nous incitent à poursuivre dans cette voie. Le nouveau programme présente 5 engagements forts et 26 mesures incitatives, avec pour ambition de s’inscrire dans la continuité du précédent et, surtout, de susciter une génération sans tabac. Je tiens à saluer ces engagements du ministère, et je ne doute pas, madame la ministre, que vous suivrez parfaitement ce programme.

visant à interdire la fabrication, la vente, la distribution et l’offre à titre gratuit des cigarettes dites puffs. Que sont ces ces cigarettes ? Les puffs – littéralement, « bouffées », en anglais – sont des cigarettes électroniques à usage unique. Commercialement présentées comme « ludiques », elles capitalisent sur un emballage coloré et sur un large panel de goûts fruités. Leur prix, qui ne s’élève guère à plus de 7 euros l’unité, complète cet arsenal attractif. Ces choix marketing ont pour cibles leurs principaux consommateurs : les jeunes. Quelques chiffres nous permettent d’en mesurer l’ampleur : 73 % des mineurs en ont déjà entendu parler ; malgré l’interdiction pénale de la vente de ces produits aux moins de 18 ans,

À ce stade, je souhaite simplement rappeler que le tabagisme est la première cause de mortalité évitable en France, qu’il cause 75 000 décès par an, que le tabac coûte à l’État plus de 1,6 milliard d’euros et qu’il représente un coût social annuel estimé à environ 160 milliards d’euros. Il y a donc urgence, mes chers collègues, à interdire ces puffs, qui peuvent constituer une porte d’entrée idéale. une porte d’entrée idéale. Une seule puff renferme 500 bouffées, soit l’équivalent d’un paquet de cigarettes entier. Il peut également contenir jusqu’à 2 % de nicotine, dont les effets sont dévastateurs pour la santé c’est une substance à la fois addictive et nocive, avec des conséquences sur le développement cérébral, comme le prouvent certaines études. L’utilisation de ces cigarettes contrevient également aux ambitions du programme national de lutte contre le tabac, dont le premier axe concerne la protection des jeunes des jeunes à l’égard du tabagisme. En effet, pour presque 1 jeune de 17 ans sur 2, les puffs constituent la première porte d’entrée dans le tabagisme. Les interdire nous offrirait donc de nouvelles marges de manœuvre pour répondre à

Leur interdiction s’avère également indispensable d’un point de vue écologique. L’Alliance contre le tabac souligne son impact environnemental majeur.

les plus énergivores de la planète, et son rejet dans les milieux naturels constitue l’une des catastrophes écologiques les plus désastreuses pour nos sols, pour nos eaux et pour la biosphère en général. Lutte contre le réchauffement climatique et consommation de puffs sont donc antinomiques.

Je terminerai mon propos en évoquant les enjeux juridiques au niveau européen. En effet, si ce texte était adopté par le Parlement, la Commission européenne devrait rendre son avis

Une exception est possible lorsque l’intention de l’État membre est justifiée par des motifs spécifiques à la situation du pays, à condition qu’il y ait un objectif de protection de la santé publique. Au niveau européen, l’Allemagne, la Belgique et l’Irlande travaillent sur des législations similaires. Ce tir groupé peut mettre la pression au niveau européen pour faire évoluer la directive sur les produits du tabac et les produits connexes. Mes chers collègues, en votant cette proposition de loi, nous agissons pour la protection de nos enfants, mais aussi de notre environnement. Le groupe Union Centriste votera donc en faveur de cette initiative parlementaire, et il remercie une nouvelle fois son rapporteur. Bravo ! La parole

les puffs représentent une nouvelle occasion d’élargir leur offre, tout en faisant entrer les utilisateurs dans l’univers de la nicotine. Même si les effets à long terme des cigarettes électroniques sur la santé ne sont pas encore totalement connus, il a été établi que les substances toxiques qu’elles généraient pouvaient provoquer des cancers et augmenter les risques de pathologies cardiaques et pulmonaires. Ces cigarettes électroniques, pensées à l’origine pour permettre la diminution, voire l’arrêt, de la

tabac. Même les puffs qui ne contiennent pas de nicotine posent un problème de santé publique, en asservissant les jeunes au geste du vapotage.

à portée de main, s’éloigne donc à grands pas. La prévalence du tabagisme quotidien chez les jeunes de 17 ans avait pourtant baissé significativement entre 2017 et 2022 – vous l’avez souligné, madame la ministre –, bien au delà des objectifs, et même au delà des

pour eux, avec des couleurs et des goûts alléchants qui donnent envie d’essayer et de renouveler l’expérience ? Ce phénomène de mode est accentué par les réseaux sociaux, puisque des influenceurs sont payés pour vanter les nouveaux goûts disponibles ou se mettre en scène avec

Le 4 décembre 2023, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité cette proposition de loi visant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique, également appelés puffs. Les industriels du tabac n’ont pas attendu le vote du Sénat pour lancer la « maxipuff », encore plus volumineuse et dangereuse puisqu’elle contient 9 000 bouffées possibles avant épuisement de la réserve, soit l’équivalent de 18 paquets de cigarettes. Reconnaissons le, l’industrie du tabac se trompe rarement en matière de marketing, à grand renfort de communication sur les réseaux sociaux. Ces vapoteuses aux couleurs vives portant des leds multicolores qui s’allument à mesure qu’on les utilise, et aux goûts toujours plus extravagants, les jeunes se les arrachent Il est bien loin le temps des cigarettes en chocolat ! Notre collègue députée Francesca Pasquini ne s’est pas trompée en déposant cette proposition de loi visant à interdire ces cigarettes électroniques jetables ou à usage unique, qui peuvent comporter de la nicotine. Dans une tribune publiée le 30 avril 2023 dans, une vingtaine de spécialistes apportaient leur soutien à cette initiative parlementaire et qualifiaient les cigarettes électroniques jetables de « fléau environnemental et sanitaire qu’il faut interdire d’urgence ». Cela

déplorables. Par ailleurs, ces cigarettes jetables sont une porte d’entrée vers la consommation de nicotine. Face à la baisse de la consommation de tabac dans notre pays, l’industrie du tabac utilise un marketing agressif pour convertir les générations à venir, au mépris de la santé publique.

Pourtant, selon l’Académie nationale de médecine, la puff « constitue un piège particulièrement sournois pour les enfants et les adolescents de ralentir, voire d’inverser [la] tendance vertueuse […] d’une quasi disparition du tabagisme en France le consensus autour de l’interdiction des puffs nécessite désormais une validation de la Commission européenne. Après le rejet par celle ci d’un projet d’interdiction des puffs en Belgique, le Gouvernement devra soutenir le présent texte et peser dans les négociations sur l’actualisation de la directive sur les produits du tabac. La sacro sainte liberté de circulation des marchandises ne doit pas primer la santé de nos jeunes.

Les commerçants de la filière nous ont également fait part de leur soutien à l’interdiction de ce produit, qui ne représente qu’une part négligeable de leurs ventes. Après une première lecture à l’Assemblée nationale, qui a voté le texte à l’unanimité, et le travail de la commission, je sais que nous trouverons à notre tour

Cela a été dit, cette proposition de loi vise un double objectif, de santé publique et écologique. D’une part, la cigarette électronique non rechargeable est le vecteur d’un marketing agressif, avec des emballages et des saveurs qui ont pour objectif de séduire une clientèle jeune. Ne nous y trompons pas : la puff n’est pas l’outil de sevrage tabagique privilégié par les fumeurs ou les anciens fumeurs. Au contraire, elle constitue une entrée vers la dépendance à la nicotine. Le nombre de consommateurs de cigarettes électroniques âgés de 17 ans a triplé en cinq ans, et la facilité d’achat et d’utilisation de ces cigarettes n’est pas dépourvue de lien avec cette recrudescence.

évidence écologique : ces produits, lorsqu’ils sont usagés, sont très peu déposés dans des points de collecte en vue de leur recyclage ; et leurs composants étant difficilement dissociables, il est La lutte contre le tabagisme est un défi pour un pays comme le nôtre, qui demeure très fumeur. Notre politique doit être claire : le vapotage peut s’envisager comme moyen de sevrage de la cigarette, mais jamais comme une porte d’entrée vers l’addiction à la nicotine. Cette proposition de loi est un premier pas pour faire du vapotage uniquement le substitut nicotinique qu’il doit être. Mais il reste du chemin à parcourir en vue de garantir la santé des utilisateurs, notamment au travers d’une meilleure réglementation encadrant les liquides vaporisés

Les liquides sans nicotine font l’objet d’une réglementation insuffisante, alors même que leur utilisation dans le cadre d’un sevrage tabagique est douteuse. Les règles en matière de promotion et d’emballage sont encore trop souvent contournées. Quant aux contrôles et aux amendes de la DGCCRF, ils sont parfois insuffisants. La filière française, qui emploie aujourd’hui entre 13 000 et 20 000 personnes, semble volontaire pour s’engager dans de tels chantiers.

Nous manquons encore de certaines données scientifiques, ce qui doit nous appeler à une certaine vigilance lors de nos arbitrages. Nous avons également la responsabilité de prévoir des moyens préventifs et éducatifs, parallèlement à cette interdiction.

; de nouveaux accessoires, stars des cours de récréation, aussi dangereux pour la santé que pour l’environnement. Emballage aux couleurs vives, lumière clignotante incluse, prix modique, produit facile à trouver

aucune mesure de contrôle de l’âge ; il suffit de cliquer sur un bouton pour affirmer que l’utilisateur est majeur. Cela me rappelle vaguement les soi disant « filtres » de certains sites interdits aux mineurs… Voilà quasiment un an, jour pour jour, j’alertai le Gouvernement sur les conséquences néfastes des puffs sur la santé de nos adolescents. N’attendons plus aussi longtemps pour légiférer lorsqu’il s’agit de la santé de nos enfants ! L’autre problème majeur que pose la puff est d’ordre environnemental. Notre jeunesse s’illustre par

enrayer le fléau du tabagisme. Lorsqu’une drogue disparaît, une autre la remplace presque immédiatement. D’autres substances, qui commencent d’ailleurs à pénétrer notre marché, doivent dès à présent faire l’objet de toute Je veux parler, par exemple, des sachets de nicotine, déjà interdits dans de nombreux pays de l’Union européenne, mais qui échappent pourtant à tout encadrement de la part du législateur français. Parce qu’il vaut mieux prévenir que guérir, n’attendons pas qu’une substance nocive devienne une habitude de consommation pour agir et pour protéger notre jeunesse. Les sénateurs Les Républicains continueront de faire barrage aux dangers qui menacent la santé de nos jeunes et la préservation de notre environnement. Madame la ministre, monsieur le rapporteur – je veux saluer votre implication et l’intérêt que vous avez porté à ces questions depuis votre arrivée au Sénat –, mes chers collègues, cette proposition de loi reçoit notre approbation au delà des clivages politiques, parce que nous avons tous à cœur de servir

Dans sa rédaction actuelle, en effet, le projet d’article L. 3513 5 1 du code de la santé publique sanctionne leur mise à disposition à titre gratuit ou onéreux. Cette sanction implique soit un constat de flagrance de la transaction du vendeur vers l’acheteur, soit la verbalisation au vu des registres de vente. L’extension que nous vous proposons permettra de sanctionner plus largement la détention de ces produits dans les réserves des magasins ou leur exposition dans les rayons, ce qui, à la fois, favorisera les constats par les agents de contrôle et permettra de viser de plus grands volumes destinés à la vente en infraction à la loi. En second lieu, l’amendement tend à permettre aux agents de la concurrence,

il dispose d’une batterie non rechargeable. Il s’agit d’anticiper l’imagination des fabricants, qui ont déjà commencé à commercialiser dans certains pays des kits

n° 3. Je vais mettre aux voix l’article 1,modifié. L’article 2 étant supprimé, le vote sur l’article 1 vaudra vote sur l’ensemble de la proposition de loi.

et du projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010 837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution La procédure accélérée a été engagée sur ces textes. Il a été décidé que ces textes feraient l’objet d’une discussion générale commune.

assemblée le projet de loi relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires. Aujourd’hui, nous sommes appelés à débattre d’un texte tout aussi crucial pour notre politique de transition énergétique : le projet de loi sur la réforme de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

des milliers de femmes et d’hommes qui exploitent ces cathédrales technologiques. Il repose surtout sur l’existence d’une organisation permettant un contrôle indépendant et reposant sur les meilleures compétences possible. Suivant les recommandations du rapport du député Jean Yves Le Déaut, en 1998, le processus d’amélioration et de réorganisation des services de l’État s’est enclenché voilà plus de vingt ans. Un établissement public sous tutelle gouvernementale résultant de la fusion de plusieurs agences et services de l’État, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), a ainsi été créé en 2002, avec déjà, à l’époque, des difficultés inhérentes à toute réforme organisationnelle. en 2006, la loi Transparence et sécurité nucléaire a permis le passage d’une direction d’administration centrale à une autorité administrative indépendante – indépendante non seulement des exploitants, mais également du Gouvernement. Ce fut la création de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), chargée du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Plus de dix sept ans après, la conclusion collective que nous pouvons en tirer est que cette organisation a été au rendez vous

Je ne vais pas entrer dans l’énumération de tous les projets associés à cette relance, qui vont accroître significativement et durablement le volume et la complexité des dossiers de sûreté et de radioprotection.

Gravelines et au Bugey. Il y a encore la relance de grands programmes de recherche et développement : développement de nouveaux réacteurs innovants et modulaires et réactivation d’un programme d’investissements dans les infrastructures du a enfin la consolidation de l’amont et de l’aval du cycle du combustible. Pour mener ces chantiers, le Gouvernement s’attache à mettre tous les maillons du nucléaire civil à leur meilleur niveau : réforme des administrations publiques, nationalisation d’EDF, mise en œuvre d’un plan Marshall des compétences, sécurisation et accélération des procédures administratives. Le Gouvernement a aussi engagé une réflexion visant à faire évoluer l’organisation de la sûreté nucléaire pour qu’elle continue de répondre au mieux à la mission d’assurer un contrôle indépendant et efficace du nucléaire civil en France, en s’inspirant, comme en 2006, des meilleurs modèles internationaux. insiste, ce projet de loi ne modifie pas d’une virgule le cadre de sûreté et de radioprotection français applicable aux exploitants.

ce qui limite l’efficacité du pilotage de leurs moyens et nécessite des dizaines de documents cadres négociés pour organiser leurs relations au quotidien. Ensuite, ces deux structures ont des processus et des outils internes distincts, ce qui limite le partage d’informations et l’efficacité des instructions et de la gestion de crise. dans le contexte de relance du nucléaire, l’ASN et l’IRSN pourraient se disputer des compétences rares similaires, limitant les synergies qu’une mise en commun offrirait dans un contexte de tension sur ces mêmes compétences. Cette réflexion s’était déjà imposée lors de l’examen du dernier texte sur le nucléaire au Parlement. Je veux le dire d’emblée, cette méthode, qui avait vu à l’époque intervenir la proposition de réforme au milieu de la navette parlementaire, n’était pas adaptée à l’enjeu,

Le texte que nous examinons aujourd’hui a fait l’objet d’un mois et demi de consultations auprès de neuf instances différentes, de dizaines de réunions de travail avec le corps social de l’ASN et de l’IRSN, d’un examen minutieux par le Conseil d’État pour en conforter la solidité juridique et élaborer une étude d’impact de deux

ni l’IRSN, mais une nouvelle Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR). Elle réunira, à compter du 1 janvier 2025, les compétences et missions des actuels ASN et IRSN. C’est un calendrier ambitieux,

augmentation des rémunérations, parcours de carrières plus larges, ou encore meilleure allocation des compétences rares de l’État. Il contribue également à la relance nucléaire, en permettant aux maîtres d’ouvrage de projets nucléaires, en particulier EDF, de passer leurs marchés selon des modalités plus adaptées à leurs contraintes industrielles et de renforcer la protection des intérêts essentiels de la Nation, afin de tenir compte de l’évolution du contexte international.

puisse faire encore progresser un texte qui nous permettra de maintenir dans la durée l’excellence de la sûreté nucléaire et de la radioprotection française, auxquelles le Gouvernement, comme tous les Français, est pleinement attaché.

nous sommes réunis aujourd’hui pour examiner le projet de loi relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, afin de répondre au défi de la relance de la filière nucléaire et du projet de loi organique associé. J’ai organisé durant les premières semaines de janvier une vingtaine d’auditions. J’ai souhaité travailler en bonne intelligence avec la commission des affaires économiques, saisie pour avis, mais aussi, pour quatre articles, au fond. Certaines de ces auditions ont été menées conjointement avec Patrick Chaize, dans un très bon climat.

Nous avions été très nombreux, au Sénat, à déplorer la méthode employée : cette proposition n’avait fait l’objet d’aucune concertation ni d’aucune évaluation et n’avait pas été soumise à la première assemblée saisie, c’est à dire le Sénat. La proposition du Gouvernement avait finalement été rejetée par les députés.

Pour l’examen de ces textes, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable s’est fixé une priorité essentielle : maintenir notre sûreté nucléaire au niveau d’exigence le plus élevé possible, tout en l’adaptant aux enjeux de la décennie actuelle et J’ai ainsi effectué une instruction à charge et à décharge, en m’appuyant notamment sur le rapport de l’Opecst et sur une étude de législation comparée demandée aux services du Sénat. Cette instruction m’a conduit à identifier cinq avantages de la refonte proposée de la gouvernance de la sûreté nucléaire. premier est une efficacité accrue. J’ai pu constater, au fil de mes auditions, que l’excellence du système français de sûreté nucléaire est reconnue par l’ensemble des parties prenantes, à l’échelle nationale comme internationale. notre système de sûreté nucléaire doit aujourd’hui s’adapter à l’évolution du flux de demandes : vous le savez, la relance du nucléaire est un chantier d’une ampleur inédite, un programme hors norme. La nouvelle organisation permettra de mettre fin aux frictions qui ont pu se produire dans les échanges entre l’ASN et l’IRSN, ainsi qu’aux différences de priorisation, qui donnent lieu aujourd’hui à des délais supplémentaires dans la prise de décision. Le deuxième avantage est une meilleure adaptation aux enjeux contemporains de la sûreté nucléaire. Le premier enjeu contemporain est celui des petits réacteurs modulaires, ou SMR, développés notamment par des start up. J’ai pu entendre, dans le cadre de mes auditions, les start up françaises, qui sont engagées dans une véritable course technologique contre les autres puissances nucléaires.

Pour assurer leurs missions en cas de crise, l’IRSN et l’ASN disposent chacun d’un centre de crise, d’une organisation spécifique et de moyens propres. En la matière, la fusion permettra aux services de l’État de disposer d’un interlocuteur unique et fluidifiera les échanges entre les différentes équipes. Le quatrième avantage est une clarification de la communication. Combien de nos concitoyens sont aujourd’hui capables de distinguer les missions de l’ASN de celles de l’IRSN ? Émanant de deux institutions différentes, la communication sur ces sujets a pu donner lieu, par le passé, à des cafouillages préjudiciables. La réforme permettra à la nouvelle autorité de parler d’une voix commune et, partant, facilitera l’identification par le public de l’autorité décisionnaire.

les paramètres retenus par le Gouvernement constitueront des outils pour rendre la future Autorité plus attractive. Une part de la nécessaire réaction face au déficit d’attractivité des instances de sûreté réside néanmoins également dans l’augmentation des rémunérations et des moyens humains, un sujet qu’il faut inscrire dans la durée que le Gouvernement n’a pas, à ce jour, voulu prendre suffisamment au sérieux, en dépit de nombreuses alertes parlementaires. Vous l’aurez compris, mes chers collègues, la réforme de la gouvernance de la sûreté nucléaire permettra de renforcer le système de sûreté nucléaire français dans un contexte hors norme.

les conclusions de l’expertise seraient orientées dans le sens de la décision ou, inversement, la décision, censée tenir compte de l’expertise, mais également d’enjeux comme l’approvisionnement en électricité du pays, pourrait ne pas être assez autonome vis à vis des avis scientifiques présentés

du projet de loi constituait un recul, sur la méthode, en renvoyant le sujet au règlement intérieur de la future Autorité, et surtout sur le fond, en prévoyant une distinction entre processus d’expertise et de décision uniquement dans le cas d’une prise de décision par le collège, ce qui concernerait 30 dossiers par an, contre 300 aujourd’hui. Un redémarrage de centrale nucléaire n’aurait ainsi plus fait l’objet d’une expertise distincte du reste de l’instruction La commission a préféré adopter une position d’équilibre, qui préserve la fluidité permise par la fusion des deux entités, tout en garantissant la confrontation des doutes indispensable à la sûreté. Le premier avantage du texte adopté en commission est qu’il étend le champ de la distinction à l’ensemble des dossiers à enjeux, au delà des 30 sujets annuels nécessitant une décision du collège. Son deuxième avantage est que nous proposons une distinction des responsabilités plutôt que des « processus notion particulièrement floue retenue dans le texte initial. On s’assurera ainsi que le signataire de l’expertise n’est pas le même que le signataire de la décision. Mais la distinction des responsabilités, donc des signataires, ne suffit pas. Notre objectif est de consacrer une distinction entre expertise et décision qui ne soit pas que de papier ; il nous a semblé que ce principe devait se traduire concrètement dans l’organisation des instructions. C’est pourquoi nous avons souhaité préciser que le règlement intérieur de l’Autorité fixera les modalités organisationnelles de distinction et d’interaction des personnels chargés de l’expertise et de la décision. Cette précision garantira, sur un dossier donné, que les personnes chargées de l’expertise, d’une part, et de la décision, d’autre part, seront bien identifiées. Notre idée n’est pas ici de recréer, au sein de l’ASNR, un pôle expertise distinct d’un pôle décision

en donnant une assise juridique forte aux groupes permanents d’experts, les GPE, comme le proposait le rapport de l’Opecst. Ces groupes, constitués de spécialistes, contribuent au processus d’expertise, en lui apportant un regard critique et des compétences spécialisées.

C’est pourquoi la commission a adopté un amendement tendant à intégrer au texte, comme le proposait le rapport de l’Opecst, le principe de publication des résultats d’expertise, pour maintenir un niveau de transparence équivalent à celui qui est atteint dans le système actuel. Le troisième risque que nous avons identifié concerne le maintien des activités de recherche. du projet de loi comportait des risques pour la conduite des activités de recherche de la future ASNR, activités qui sont le socle de l’expertise en matière de sûreté et de radioprotection. Les acquis de l’IRSN, sa notoriété et sa visibilité dans le monde de la recherche devront être préservés, comme l’a souligné le rapport de l’Opecst. En particulier, l’ASNR devra poursuivre la collaboration engagée par l’IRSN avec les industriels du secteur nucléaire, collaboration indispensable à la recherche en sûreté nucléaire. le quatrième risque du texte initial était relatif à l’association du Parlement et de la société civile. De nombreux sujets majeurs seront renvoyés au règlement intérieur de la future autorité. Ce choix est justifié par la nécessité d’assurer une plus grande souplesse dans le fonctionnement de l’Autorité.

(Anccli) et les commissions permanentes compétentes des deux assemblées. En définitive, le projet de loi que nous examinons aujourd’hui est un texte rééquilibré, qui adapte la sûreté nucléaire aux enjeux de notre décennie, tout en maintenant la sûreté nucléaire au niveau d’exigence, mais aussi de transparence, le plus élevé possible.

les projets de loi ordinaire et organique que nous examinons aujourd’hui procèdent à trois réformes techniques, destinées à accompagner la relance de la filière française du nucléaire, actée par la loi du 22 juin 2023, La commission des affaires économiques a été chargée de l’examen au fond des articles 12 et 16 à 18 du projet de loi ordinaire, c’est à dire de ceux qui portent sur la simplification des règles de la commande publique, ainsi que sur le repositionnement du haut commissaire à l’énergie atomique Elle s’est saisie pour avis des autres articles des deux projets de loi, relatifs à la création de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Lors de l’examen de la loi Nouveau nucléaire, le Gouvernement avait déposé à l’Assemblée nationale deux amendements tendant à fusionner l’Autorité de sûreté nucléaire et l’Institut de radioprotection et de

En rejetant ces amendements présentés par le Gouvernement à la hâte – vous l’avez vous même reconnu, monsieur le ministre –, après le vote massif du Sénat sur ce texte, notre commission s’était opposée à une réforme mal anticipée et mal évaluée. En saisissant l’Opecst, elle avait remis les parlementaires au cœur des enjeux. Le nouveau projet de réforme est plus abouti ; nous pouvons néanmoins regretter que nous n’ayons pu auditionner le ministre chargé de ce dossier. Il est plus abouti, disais je, car il est le fruit du rapport de l’Opecst, d’une dizaine de consultations et d’un an de concertation. Il arrive à un moment crucial de la relance du nucléaire, le Gouvernement devant proposer de nouvelles régulations et programmations énergétiques, dans le projet de loi relatif à la souveraineté énergétique, ainsi que dans le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie. Notre commission soutient aujourd’hui, dans son principe, le nouveau projet de réforme, plus abouti que le précédent. Parce qu’il vise à fluidifier les procédures d’instruction, à sûreté inchangée, il est indispensable à la relance du nucléaire. À l’heure où les dossiers vont se multiplier, renforcer l’efficacité du système n’a rien de superflu. Certes, les modalités du projet posent des défis en matière de continuité des procédures, de valorisation des compétences et de maintien des standards. Pour autant, à terme, le projet est de nature à renforcer la confiance du public, car l’ASNR sera une autorité administrative indépendante, Dans le cadre de mes travaux préparatoires, j’ai entendu une quarantaine de personnalités, au cours d’une vingtaine d’auditions. Au total, j’ai proposé à notre commission 37 amendements, selon quatre axes consolider la gouvernance de la filière du nucléaire, simplifier les règles de la commande publique, faire suite aux travaux de la loi Nouveau nucléaire et conforter l’organisation de l’ASNR. Déjà, 25 de ces amendements ont été adoptés en commission ; j’aurai l’occasion de revenir sur les autres, qui vous seront soumis Le premier axe de mes travaux a pour objet de consolider la gouvernance de la filière nucléaire, en renforçant les attributions et le fonctionnement du HCEA et en prévoyant que le Parlement puisse le saisir pour avis et se prononcer sur sa désignation. ans après sa création par le général de Gaulle, faire du HCEA la vigie de la relance du nucléaire. Le deuxième axe vise à simplifier les règles de la commande publique pour les projets nucléaires, en confortant les dérogations prévues en matière d’allotissement, de durée des accords cadres et de règles de publicité et de concurrence, et en ajoutant un critère de crédibilité et une possibilité d’avenant. Ces souplesses sont nécessaires pour prévenir tout risque d’interface, de rupture et,, de surcoût.

en proposant d’appliquer les recommandations du rapport de l’Opecst et de réintroduire des dispositions instaurant une règle de parité, dans le collège de l’autorité, et une règle de publicité, dans sa commission des sanctions. C’est un gage de cohérence. travail vise enfin à conforter l’organisation de l’ASNR, notamment en matière de garantie d’indépendance et de déontologie, de séparation entre les processus d’expertise et de contrôle, de publication des rapports et des décisions, ou d’association de l’Opecst et des commissions permanentes. Je souhaite aussi consacrer l’indépendance de l’Autorité et sanctuariser ses activités régaliennes. Je veux, à ce stade de notre débat, remercier le rapporteur Pascal Martin de nos échanges constructifs.

s’était engagée dans le nucléaire sans qu’à aucun moment le Parlement se soit prononcé sur les choix scientifiques lourds et de long terme que cela impliquait. Depuis sa création il y a quarante ans, l’Opecst, que j’ai l’honneur de présider, s’intéresse de près au sujet majeur de la sûreté nucléaire dans notre pays.

Tirant les conséquences de l’accident de Tchernobyl, ce rapport avait comme principale recommandation la création d’une « agence nationale de la sécurité et de l’information nucléaires », indépendante des pouvoirs publics et des exploitants d’installations nucléaires, autrement dit la future ASN.

L’analyse des systèmes étrangers, loin d’être tous identiques, avait également convaincu nos prédécesseurs. Il a néanmoins fallu attendre dix neuf longues années avant que cette nouvelle organisation ne se mette en place, ce qui ne s’est pas fait sans remous ni polémiques. La nouvelle étape proposée aujourd’hui par le Gouvernement me conduit à faire trois séries d’observations. Premièrement, sur la forme, je me félicite que cette réforme soit entreprise au travers d’un projet de loi spécifique, après la maladroite tentative de l’an dernier par amendement gouvernemental de dernière minute. La sûreté de nos installations nucléaires est un impératif absolu, sur lequel le Parlement doit pouvoir prendre le temps de débattre. Dès le printemps dernier, l’Opecst a organisé une audition publique réunissant toutes les parties prenantes pour faire un point sur les enjeux et les éventuelles conséquences de la réforme. Puis, sur saisine de la commission des affaires économiques du Sénat, alors présidée par Sophie Primas, avec mon collègue député Jean Luc Fugit, nous avons mené de nombreuses auditions pour évaluer en profondeur les impacts d’une réorganisation de l’ASN et de l’IRSN. Notre rapport, adopté par l’Office en juillet dernier, contenait 17 recommandations, qui ont inspiré, au moins en partie, le travail des deux commissions du Sénat sur le projet de loi. Ma deuxième série d’observations porte sur le contexte de la réforme. Nous ne pouvons plus raisonner aujourd’hui comme nous le faisions au début des années 2000, période de grand calme dans le domaine nucléaire. La relance du nucléaire, avec la construction de nouveaux réacteurs, l’arrivée de petits réacteurs innovants, l’adaptation au changement climatique, la prise en compte de la menace cyber, sans oublier le suivi du parc actuel et du démantèlement d’installations anciennes, nécessitent que l’organisation du contrôle de la sûreté soit renforcée et robuste. Il est important de s’en préoccuper sans perdre de temps et d’anticiper la charge des années à venir. Cette nouvelle donne, inédite par son ampleur, doit être prise en compte. Elle représentera un immense défi pour la nouvelle ASNR.

qui a détecté le problème de corrosion sous contrainte dans un certain nombre de ses réacteurs, avant d’engager un dialogue technique avec l’IRSN et l’ASN. La sûreté nucléaire est une « fabrication quotidienne », faite de discussions entre l’exploitant, les experts et l’autorité de sûreté. De même, l’expertise est multiple : elle existe chez l’exploitant, au sein de l’IRSN, bien sûr, à l’ASN, mais aussi au sein des groupes permanents d’experts, qui ont un rôle clé pour certains sujets particulièrement sensibles.

L’Office tient à ce qu’un haut niveau d’information se maintienne, voire se renforce, grâce à l’utilisation de tous les canaux de diffusion possibles. Car, si l’acceptabilité du nucléaire passe par un niveau de sûreté élevé, elle dépend aussi d’une très grande transparence. L’Office a pleine confiance dans les acteurs actuels de la sûreté nucléaire et dans leur capacité à réussir la réforme aujourd’hui proposée. Monsieur le ministre, cette responsabilité vous incombe également,

Je n’en suis pas coutumier, tant je considère – je sais que nous sommes nombreux dans cet hémicycle à partager cette conviction – que notre mission est de légiférer, de discuter et d’améliorer les textes de loi, et non pas de refuser le débat. Une question préalable n’est justifiable que si elle répond à plusieurs difficultés. La première, bien sûr, est l’importance du sujet. Sommes nous ici face à un enjeu majeur pour la sécurité nationale ? La réponse est bien évidemment oui Quand on est, encore aujourd’hui, le deuxième pays le plus équipé du monde en centrales nucléaires, qui plus est des centrales vieillissantes ou, pour la dernière, en rodage de très longue durée, sûreté et sécurité nucléaires sont non pas de petits sujets, mais des questions essentielles pour l’avenir du pays. La seconde difficulté tient évidemment au temps et aux moyens réservés au débat parlementaire. Avons nous eu ce temps ? La réponse est à l’évidence non ! J’ai même le sentiment qu’il y a consensus sur ce point.

mais il convenait dans ce cas de repousser l’examen de ce projet de loi. Le temps politique, légitime, de la constitution d’un casting gouvernemental ne pouvait en aucune manière passer avant la sécurité collective des Français.

que vous faites du mot de « responsabilité » : est ce vraiment responsable d’accélérer après avoir fait le constat qu’il n’y avait pas eu débat ? Il y a là une contradiction sur laquelle il nous faudra revenir.

si fiers, y compris sur les bancs de la majorité sénatoriale ! Nombre de questions restent donc sans réponse. Certes, un mot magique s’est imposé : « fluidité C’est fou à quel point, dès qu’il s’agit du nucléaire, il faut des mots magiques ! Abracadabra, et d’un coup de baguette magique l’État fait disparaître l’IRSN ! Par parenthèse, je ne sais pas si c’est avec la même formule, mais il a aussi fait disparaître entre temps la fée qui tenait la baguette

réacteurs, sans oublier le stockage des déchets et la multiplication des projets de petits réacteurs modulaires, aux technologies aussi complexes que différentes suivant les producteurs.

les équipes de l’ASN et de l’IRSN seront probablement soumises à une très forte pression pour assurer l’instruction des dossiers dans des délais aussi courts que possible. » Tout est dit ! On l’aura donc compris, l’ASN a besoin de monde pour assurer ses propres missions et lorgne par conséquent le personnel de l’IRSN, bien plus étoffé.

Les analyses réalisées par le sociologue spécialisé en analyse de risque Charles Perrow sur l’accident nucléaire de Three Mile Island, aux États Unis, le 28 mars 1979, et sur d’autres accidents dans les secteurs aéronautique, pétrochimique et maritime concluent au fait que la multiplicité et la variété des points de vue permettent d’assurer un “scepticisme organisé”, le contraire d’une confiance aveugle, et améliorent significativement le niveau de sûreté en évitant le monolithisme de l’organisation. »

souvent cités, ont certes une structure unique, mais aussi des laboratoires de recherche indépendants dans les grandes universités, qui jouent ce rôle de recul, voire de poil à gratter. J’ai donc une question simple à vous poser, monsieur le ministre prévoyez vous d’accorder des budgets spécifiques à des universités françaises, pour qu’elles puissent, en toute autonomie, se poser des questions relatives à la sûreté et à la sécurité nucléaires ? Voilà une question intéressante, parmi d’autres, dont nous n’avons pu débattre. Nous partageons avec le rapporteur Pascal Martin, dont je salue le travail réalisé dans l’urgence, une certaine culture du risque. Je fus longtemps vice président de Nantes Métropole chargé du risque. Nous connaissons ces exercices où l’on imagine l’inimaginable avec des chercheurs en sciences sociales ou de simples citoyens ; ces moments sont essentiels, car ils suscitent des questions que l’on ne s’était pas posées. Nous pouvons craindre la fin, ou à tout le moins l’affaiblissement, de ces regards extérieurs et de cette triangulation qui est le socle de la sécurité et de la sûreté.

certains des amendements de suppression du Gouvernement sont sur ce point extrêmement inquiétants, confirmant notre inquiétude sur la vraie raison de cette fusion : accélérer, toujours accélérer, quitte à réduire la sécurité.

car ils estiment qu’au lieu d’accélérer le retour du nucléaire, elle constituera l’un des éléments des futurs blocages. Je n’ai pas le temps, même en dix minutes, d’énumérer tous les avis selon lesquels cette réforme est précipitée,

Je ne vois pas en quoi le passage d’un système dual à un système unique remettrait gravement en cause notre système de sûreté nucléaire et de radioprotection, comme cela a été avancé. De nombreux pays dans le monde – les États Unis ou le Canada, par exemple – disposent d’un système unique est ce à dire que le niveau de protection de la population et de l’environnement y est plus faible qu’en France ? Certes, des risques sont associés à cette réforme – je ne le nie pas, je l’ai d’ailleurs toujours dit –, mais je pense que nous y avons apporté des réponses fortes par les amendements adoptés en commission, notamment en matière de distinction entre l’expertise et la décision.

Il serait donc tentant de renoncer à la réforme, pour ne pas déstabiliser le système. Toutefois, la pression continuera de s’amplifier dans les années à venir, et il sera alors trop tard pour bénéficier des avantages attendus de la réforme. les auteurs du rapport de l’Opecst, au regard du calendrier de travail, une fenêtre d’opportunité s’offre au législateur, mais elle pourrait rapidement se refermer : s’il faut agir, il faut le faire dès à présent. vous affirmez que ce qui manque aujourd’hui, ce sont les vocations, les ressources humaines et les moyens alloués à l’expertise comme au contrôle. Je vous rejoins sur ce point. Reste que l’augmentation des rémunérations et des moyens humains ne relève pas d’une loi ordinaire. Par ailleurs, je considère que la nouvelle organisation permettra justement d’éviter la dispersion des compétences techniques et scientifiques rares, ce que des mesures budgétaires et salariales ne pourront pas faire seules. Je regrette également que nous n’ayons pu entendre un ministre sur ce texte.

Je dois dire à Ronan Dantec que, même si nous avions eu six mois de plus pour discuter du sujet, sa position n’aurait pas changé. Je lui reconnais l’honnêteté intellectuelle d’utiliser tous les moyens pour faire en sorte de stopper la relance du nucléaire, à laquelle il ne croit pas.

Ce projet de création d’une autorité de sûreté nucléaire de radioprotection est insuffisamment fondé en raison. Les objectifs, le plan de charge, les principes éthiques et déontologiques de fonctionnement des processus scientifiques et techniques, comme les perspectives de gestion des personnels et des carrières, ne permettent pas d’apporter au législateur les garanties nécessaires. Tous les organismes et parties prenantes amenés à s’exprimer sur la genèse de ce projet ont émis doutes et réserves. C’est le cas du CNTE et de l’Anccli pour les territoires les plus directement concernés. Il en est de même pour les personnels des deux établissements, dont je salue les représentants

puisque nous restons toujours dans l’attente d’un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’énergie. La politique nucléaire française devra aussi très vite intégrer la problématique de la sûreté et de la radioprotection dans le cadre d’un mix énergétique intégrant probablement les technologies nucléaires à venir – ce n’est pas rien. En définitive, et c’est le point majeur, la confiance de la population française dans la sûreté nucléaire nécessite un débat approfondi avec le grand public et l’ensemble des parties prenantes. À cet égard, il n’y aura pas de confiance sans transparence. Pour

propose de renvoyer le débat en commission, c’est pour une raison simple, qui transcende les positions entre les tenants de la filière nucléaire et ses opposants.

En effet, ce projet de loi souffre non seulement d’une méthode hâtive, mais aussi d’un objectif hasardeux. Un an après la tentative de cavalier législatif du Gouvernement, alors que nous devons entamer aujourd’hui nos débats dans l’hémicycle, aucun diagnostic,

Qui plus est, alors qu’un dialogue avait été amorcé avec l’ancienne ministre de la transition énergétique Agnès Pannier Runacher et son équipe, celui ci a été soudainement interrompu par le remaniement ministériel, qui a été pour l’énergie synonyme de dissolution du ministère de plein exercice dont la filière bénéficiait jusqu’alors.

Le point d’orgue de cette méthodologie hâtive étant l’absence d’audition ministérielle devant les commissions de l’aménagement du territoire et du développement durable et des affaires économiques,

Plus largement, notre pays reste en attente d’une loi de programmation sur l’énergie et le climat, qui devra fixer les grands objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie et de la stratégie nationale bas carbone (SNBC) et permettra de bâtir la stratégie française pour l’énergie et le climat. Cette loi de programmation, sans cesse reportée, aurait dû être adoptée avant le 1 juillet 2023. Le Gouvernement esquive une fois de plus le grand débat autour de la loi de programmation sur l’énergie et le climat, qui devrait pourtant être un préalable de la politique énergétique de la France. N’oublions pas que la Charte de l’environnement inscrite dans le préambule de la Constitution prévoit que les Français ont à connaître et doivent pouvoir discuter des politiques énergétiques et climatiques qui conditionneront la durabilité et la viabilité du monde de demain. Pour en revenir à l’objet même du texte, il n’est pas question de remettre en cause la volonté légitime de réexaminer les forces et les faiblesses de notre modèle historique de gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Il s’agit toutefois de ne pas se laisser dicter notre conduite par la précipitation, car celle ci pourrait être dommageable à bien des égards à un moment où les enjeux de la filière demandent plus que jamais de la stabilité, de la confiance et de la transparence. dommageable, tout d’abord, au regard du manque d’acceptabilité de la part des acteurs de la filière eux mêmes. Les employés de l’ASN et de l’IRSN déplorent le manque de ressources et considèrent à raison que la fusion n’apportera pas de réponse à ce problème. L’IRSN a subi une vague de démissions inédite à la suite de l’annonce du projet de fusion, et les difficultés de recrutement pèsent désormais lourdement sur l’établissement. Le risque à terme a trait à la perte des compétences pourtant indispensables à la relance de la filière. Il faut saluer l’engagement quotidien de ces femmes et de ces hommes au service de l’excellence de la filière électronucléaire française. Elle pourrait être dommageable ensuite au regard des externalités négatives de l’optimisation d’interface entre l’ASN et l’IRSN, au détriment d’autres interfaces tout aussi essentielles. La fusion annonce par ailleurs la fin de la complémentarité entre la modélisation et la mesure, pourtant essentielle dans le cadre de l’expertise en situation d’urgence et post accidentelle. dommageable, enfin, puisque l’ASNR ne garantirait pas la séparation entre l’expertise et la décision, fondement de l’intégrité du système de contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection depuis 1973, date de la création du service central de sûreté des installations nucléaires. Cette distinction est pourtant primordiale pour conforter les décisions et accroître la confiance du public. Il ne faut pas croire que les acteurs qui se battent corps et âme pour le retrait du projet de loi ne souhaitent pas l’optimisation de la gouvernante de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Bien au contraire, ils sont force de propositions, et celles ci pourraient d’ores et déjà se réaliser sans prendre le risque d’une telle réforme. La fluidité a déjà été largement améliorée ces dernières années. En témoigne le fait qu’EDF, l’IRSN et l’ASN ont d’ores et déjà défini des stratégies communes d’expertise anticipée pour l’EPR2 et les SMR, afin de sécuriser les projets, avec un cahier des charges très détaillé sur les sujets à expertiser, le cadencement et le calendrier. Autant dire que les deux institutions cherchent sans cesse à optimiser leurs interactions et que le système dual ne semble pas les entraver le moins du monde. Ce que ne veulent pas les acteurs qui s’opposent à ce projet, c’est céder à l’injonction de l’accélération, et cela pour une raison bien bien raisonnable : le risque de la déstabilisation d’un édifice, dont l’efficacité n’est plus à prouver au moment, où nous en avons le plus besoin. Il est en effet étonnant d’espérer des résultats rapides dans le cadre d’une relance de grande ampleur, au travers d’une stratégie impliquant une période significative de perturbations et de difficultés assurées dans les phases ultérieures propres aux processus de fusion. N’oublions pas que, en 2014 déjà, la Cour des comptes concluait sans ambiguïté que « la fusion des deux organismes constituerait une réponse inappropriée, par les multiples difficultés juridiques, sociales, budgétaires et matérielles qu’elle soulèverait Il est utile de garder à l’esprit à chaque instant de nos échanges la quantité d’avis défavorables au projet de loi qui émanent d’institutions scientifiques et techniques, d’organismes administratifs, de juridictions financières, et j’en passe, avis qui méritent d’être entendus à l’occasion de ce débat parlementaire. Je tâcherai de n’en citer que quelques uns, mais je vous invite sincèrement à les écouter avec intérêt avant le scrutin public solennel de mardi prochain, mes chers collègues, si vous décidez de ne pas renvoyer le débat en commission dès à présent.

L’Association nationale des comités et commissions locales d’information (Anccli), qui fédère les expériences et les attentes des trente cinq comités et commissions locales d’information, craint une précipitation quand les enjeux demandent de la stabilité et de la confiance. Elle s’inquiète tout particulièrement du manque de garanties de transparence du nouveau système de gouvernance, alors même que la participation du public est indispensable à la confiance des populations. Le Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire déplore « la la méthode par laquelle cette réforme de la sûreté nucléaire avait été introduite lors de l’élaboration de la loi du 22 juin 2023 » et s’inquiète que le projet de loi ne confirme pas les objectifs de garanties de la transparence et de l’accès aux informations tout au long du processus de prise de décision. La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement (CNDASPE) regrette quant à elle que la définition des conditions nécessaires à l’indépendance entre expertise et décision soit confiée au seul règlement intérieur, ne garantissant pas « un statut juridique solide ce que nous souhaitons, c’est assurer un dialogue plus apaisé, construit et efficace. C’est nous assurer que la marche à suivre est celle qui nous mènera bel et bien vers une relance acceptée et ambitieuse de la filière nucléaire. Pour cela, il nous semble que la seule voie envisageable est celle d’une décision nourrie par l’apport d’un temps de réflexion préalable impliquant l’ensemble des acteurs concernés par la relance du nucléaire, de la population des territoires modelés par l’industrie nucléaire jusqu’aux équipes des établissements dédiés à la sécurité et à la sûreté nucléaire, en passant par les comités et commissions locales d’information. Ainsi, mes chers collègues, au regard de la multitude des avis négatifs formulés à l’égard de ce projet de loi, de ses conséquences non maîtrisées et des lacunes manifestes dans les différents scénarios expertisés, singulièrement sur le renforcement du système dual, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vous demande d’approuver son renvoi en commission. Y a t il

Il est en effet indispensable qu’ait lieu dans cet hémicycle un débat sur la stratégie française pour l’énergie et le climat. Toutefois, quel rapport avec le texte que nous étudions aujourd’hui ?

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, pour réussir notre transition énergétique et nous passer des énergies fossiles, il nous faut de l’électricité, beaucoup d’électricité. Même pour obtenir de l’hydrogène vert ou des biocarburants, il faut de l’électricité. Si nous attendons toujours l’examen de la loi structurante de programmation énergétique, l’accélération de la production nucléaire est, en revanche, lancée. nous aurons besoin du nucléaire pour faire face aux défis qui nous attendent dans un contexte géopolitique et climatique de plus en plus incertain. L’énergie nucléaire représente un défi organisationnel et humain autant que technique, procédural et financier. Notre système repose sur quatre piliers assurant un équilibre solide, qui s’est construit tout au long de notre histoire nucléaire.

Il a été décidé de valoriser la démonstration permanente de la sûreté nucléaire s’appuyant sur le débat scientifique contradictoire autour du risque et rendu indépendant du pouvoir politique.

Pour autant, aujourd’hui, avec le développement d’internet, nous sommes dans une société de réseaux sociaux et de désinformation permanente où tous les moyens de semer le doute et d’anéantir la confiance sont en place. Je le rappelle, la confiance passe par la meilleure transparence possible. Si l’expertise ne doit pas dicter la décision, cette dernière ne doit pas étouffer la transparence de l’expertise. Or cette réforme instille le doute et affaiblit la confiance. Avec cette fusion, le Gouvernement scie le quatrième pied de la chaise sur laquelle est assise l’acceptabilité du nucléaire au moment de sa montée en puissance. La création de l’IRSN et le statut d’autorité administrative indépendante pour l’ASN reposaient sur trois exigences : la transparence, la nécessité d’éclairer les décisions publiques en matière de risques nucléaires et radiologiques et l’indépendance de la décision publique. Une quatrième exigence essentielle propre à l’environnement nucléaire français consiste en un équilibre entre la sûreté « réglée », c’est à dire la capacité à respecter les règles et à démontrer la conformité à celles ci, propre à l’ASN, et la sûreté « gérée », c’est à dire la capacité à assurer la sûreté dans toutes les circonstances, même imprévues ou imprévisibles, propre à l’IRSN. Cet équilibre ne peut pas être prescrit, mais résulte des choix organisationnels. Ce double débat peut donner une impression de complexité du système. Il est pourtant indispensable

L’étude d’impact n’apporte aucune réponse, ni sur les éventuels dysfonctionnements actuels ni sur les améliorations apportées par la nouvelle organisation. Nous relançons le nucléaire, prolongeons des réacteurs, acceptons l’arrivée de réacteurs modulaires dans un contexte de changement climatique et d’instabilité géopolitique. Dans le même temps, nous déstabilisons tout notre système de sûreté et sécurité pour aller plus vite. Mais aller plus vite vers quoi ? L’accident ? L’organisation proposée par ce texte entraînera des contre performances qui ne pourront être appréciées que dans la durée. Elles concerneront, tout d’abord, la viabilité de notre capacité de recherche, ensuite, la proportionnalité des mesures de sûreté,

Le projet de loi met également en péril à court terme notre organisation. Il fragilise les équipes dans un contexte clé de relance du nucléaire. La fusion conduira à un choc culturel. Il déconnecte la sûreté nucléaire de la sécurité nucléaire, alors que les deux sont intimement liés. Il réduit la transparence au bon vouloir de la nouvelle structure, qui opérera ses propres choix de publication. Il renvoie l’essentiel à un futur règlement intérieur, qui ne dit rien de l’équilibre organisationnel. Le calendrier esquissé de construction de la nouvelle génération de réacteurs nucléaires laisse largement

Elle devait aussi être adoptée sans examen par le Sénat, puisque les deux amendements présentés par le Gouvernement l’ont été devant l’Assemblée nationale, alors que le Sénat s’était, pour sa part, déjà prononcé. Fort heureusement, ces amendements ont été rejetés par l’Assemblée nationale et n’ont pas été réintroduits en commission mixte paritaire. Résultat, la loi promulguée au mois de juin dernier ne comporte aucune disposition relative à cette fusion. Quelle urgence justifiait une réforme aussi mal engagée ? La semaine dernière, dans son discours de politique générale, le Premier ministre Gabriel Attal a réaffirmé le rôle primordial du Sénat et rappelé qu’il n’y a pas de République sans bicamérisme. Pouvons nous en conclure que ce type de pratique ne se reproduira plus ? Quoi qu’il en soit, le refus du Parlement a donné le temps de la réflexion – il en faut. Deux projets de loi, l’un organique et le second ordinaire, proposant trois réformes techniques, ont finalement été déposés. déposés. Ils ont fait l’objet d’une étude d’impact, d’un avis du Conseil d’État et même, depuis plusieurs semaines, d’un examen par le Sénat. Il ne s’agit plus seulement de fusionner l’ASN et l’IRSN, mais de simplifier les règles de la commande publique applicables aux projets de production,

qui a saisi l’Office dès le mois d’avril 2023. Il ne faut pas s’y tromper, l’enjeu de ce texte est bien la sûreté nucléaire. Comme l’a très justement rappelé Michaël Mangeon, historien du nucléaire, devant l’Opecst, l’histoire nous montre que le système et son fonctionnement sont une cause profonde d’accident nucléaire. […] En conséquence, toute décision de réforme du système a un impact, direct ou indirect, sur la sûreté nucléaire et doit être analysée en profondeur. La réforme proposée consiste notamment à fusionner l’IRSN, établissement public industriel et commercial (Épic) chargé d’effectuer les recherches sur les risques liés à la radioactivité, qui compte plus de 1 700 agents, et l’ASN, gendarme du nucléaire, autorité administrative indépendante chargée du contrôle de la sûreté nucléaire des contrôles, des recommandations et des avis, qui compte environ 500 agents.

Cette fusion suscite des inquiétudes légitimes sur le risque de désorganisation, de perte des compétences, d’augmentation des coûts, de confusion des missions, de dégradation de l’évaluation des risques ou encore de perte de transparence vis à vis du public. Si le système actuel a donné satisfaction, cette réforme est justifiée par les perspectives de développement du nucléaire, inégalées depuis le plan Messmer, et par la nécessité de faire face aux enjeux majeurs de souveraineté énergétique. Son objectif est de fluidifier les processus à un niveau inchangé de sûreté nucléaire. L’Opecst a confirmé l’opportunité d’une telle fusion et formulé diverses recommandations ; la plupart ont été reprises par nos rapporteurs, Pascal Martin et Patrick Chaize, dont je salue le travail. C’est donc une réforme consolidée qui nous est soumise. Si elle est correctement mise en œuvre, les avantages de cette fusion seront multiples : efficacité accrue, meilleure adaptation aux enjeux contemporains de la sûreté nucléaire, amélioration de la gestion de crise, ou encore renforcement de l’attractivité. Plusieurs points mériteront une vigilance particulière, et nous aurons l’occasion de les évoquer. Sans augmentation significative des effectifs affectés aux activités de sûreté nucléaire civile et de radioprotection, tant en matière de contrôle et d’expertise que de recherche, cette fusion

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le développement et le déploiement de nouvelles structures électronucléaires constituent une ardente obligation pour assurer à la France son indépendance, sa souveraineté et une croissance respectueuse de l’environnement. Le texte qui nous est présenté, sous son aspect fortement technique, témoigne d’une volonté renouvelée d’investir dans nos centrales nucléaires. Nous ne pouvons que nous féliciter de cette victoire idéologique. Pendant des décennies, nous avons défendu, seuls ou presque, le maintien de notre puissance nucléaire, au milieu des thuriféraires de la décroissance et des pourfendeurs européens du nucléaire, soutiens, en fait, du charbon. La réunion des deux autorités que sont l’ASN et l’IRSN a provoqué, nous le savons, des inquiétudes, tant à l’Assemblée nationale qu’auprès des professionnels de la gouvernance du nucléaire.

Le travail de qualité du Sénat a permis de rendre ce texte plus lisible, d’améliorer la publicité des rapports et des communications qui seront données par la nouvelle agence et de garantir la qualité de l’expertise donnée et la célérité des autorisations transmises. Néanmoins, nous exprimons notre inquiétude devant une bureaucratisation tendancielle de notre industrie nucléaire. Ce texte devra, en pratique, atteindre l’objectif d’amélioration de la rapidité des délivrances d’autorisation de construction ou de renouvellement des centrales. Si la sécurité doit être une priorité, bien évidemment, prudence ne doit pas rimer avec impotence. Notre parc électronucléaire a été construit sans l’existence de ce dualisme d’instances, qui a, ces dernières années, contribué à affaiblir la confiance des Français envers leurs centrales nucléaires et à ralentir le processus de croissance industrielle et de création de nouvelles centrales. Depuis l’accident nucléaire de Fukushima, les activistes antinucléaires ont répandu une désinformation irresponsable sur cette source d’énergie pourtant propre, souveraine et bon marché. Ce travail lancinant a porté ses fruits empoisonnés, particulièrement auprès de notre jeunesse et au sein des gouvernements qui se sont succédé depuis lors. Résultat, notre filière nucléaire a été considérablement affaiblie et fragilisée, ce qui a mis en péril la stabilité de notre production électrique et participé à alourdir sans cesse les factures des ménages et des entreprises. Depuis sept ans, le Gouvernement a multiplié les atermoiements autour de la filière nucléaire, annonçant, dans un premier temps, sa volonté d’abaisser à 50 % la part de cette dernière dans le mix énergétique, avant de revenir sur ses décisions et d’entreprendre, bien des années trop tard, un plan d’accélération et de renouvellement de notre parc, encore largement insuffisant. sans surprise, nous soutiendrons ce texte et voterons tous les amendements visant à l’améliorer, tout en conservant son principe premier d’une autorité unique, placée sous le regard des chambres et des Français, pour garantir la sûreté de notre parc électronucléaire

L’essentielle souveraineté européenne pourrait donc, bien malgré elle, se retrouver prise en étau entre l’extrême droite américaine et certaines forces de l’extrême droite européenne. Quels que soient les résultats de ces élections, et comme l’ont prouvé les deux dernières années, notre souveraineté passe par notre indépendance énergétique. Je tiens donc à saluer la volonté de relance de la filière nucléaire manifestée par

Beaucoup ont déjà été énoncés, mais il n’est pas inutile de les citer encore. Je parle bien sûr du nouveau nucléaire, des SMR, de notre parc vieillissant, de l’indispensable adaptation au dérèglement climatique ou encore de la sécurité du marché de l’électricité, qui est un enjeu économique et géopolitique nous évoquions encore récemment dans cet hémicycle sa réforme, que nous souhaitons quasiment tous. Les enjeux sont immenses ; les réponses doivent l’être tout autant. Je salue donc le travail qui a été fourni au sein des deux commissions saisies. En

permanents d’experts devraient renforcer l’architecture de l’ASNR, et ainsi rassurer. Je crois en l’importance d’un dialogue constant entre la nouvelle ASNR et la filière nucléaire, où la recherche et l’innovation sont importantes. Il faudra néanmoins être attentifs aux conflits d’intérêts, et je pense que les dispositions de l’article 2, notamment, participent à notre vigilance.

Les missions et attributions de l’ASNR seront déterminantes, tout comme son règlement intérieur. Après les discussions en commissions, au vu des amendements déposés et des premières interventions, je n’ai aucun doute : ce sujet fera partie des plus discutés. Il sera la clé de la réussite de l’ASNR, et je forme le vœu

évoqué les salariés et leurs compétences. Les conditions du transfert des salariés, leur rémunération et les conditions d’accès à l’emploi ont un impact déterminant sur l’attractivité de ces métiers d’excellence. Nous relançons le nucléaire et avons la chance de pouvoir compter sur un vivier de personnes compétentes. Il faut leur permettre de rester en France servir notre pays, et de continuer à faire évoluer leurs compétences : les voir partir au service de puissances étrangères serait un échec majeur de cette réforme. Je terminerai en rappelant que nous avons besoin d’accorder les moyens nécessaires au secteur nucléaire. nucléaire. Ce projet de loi est une facette non négligeable de la reconstruction de l’indépendance énergétique amorcée en France et en Europe. C’est pourquoi, malgré les points de vigilance que

Madame la présidente, monsieur le ministre,

En effet, cette réforme posait de nombreuses questions, qui ne pouvaient trouver de réponses satisfaisantes dans les délais qui nous étaient impartis. Heureusement, le Gouvernement nous a écoutés, permis aux parlementaires de mieux examiner la pertinence de cette réforme, sa faisabilité, ses limites et le calendrier à suivre si l’on choisissait de la mener à terme.

construction de nouveaux réacteurs EPR de seconde génération, évolutions technologiques, prolongation de la vie des réacteurs existants, gestion des déchets nucléaires, adaptation des infrastructures au changement climatique et aux risques cyber, démantèlement des centrales en fin de vie… Autant de défis auxquels peuvent s’ajouter des imprévus, tels que les problèmes de corrosion sous contrainte rencontrés récemment dans notre parc. Avec le recul, ce contexte semble plaider efficacement en faveur d’une seule entité, issue d’un rapprochement entre IRSN et ASN. Nous voilà donc prêts à débattre de cette fusion, un an après un an après son annonce initiale, ayant pris à cœur le conseil de l’Opecst sur la nécessité de tenir un calendrier resserré de mise en œuvre de la réforme. De son côté, le Gouvernement a profité de ce délai pour affiner sa copie, désormais étayée par une étude d’impact bienvenue. Le texte établit l’ASNR en interlocuteur unique et indépendant, chargé du contrôle et de l’instruction des dossiers de sûreté et de radioprotection, ouvert sur la société, doté de moyens internes forts tout en ayant la faculté de les compléter auprès de partenaires externes et pouvant s’appuyer à la fois sur une recherche de renommée internationale et sur des groupes permanents d’experts, propices à la confrontation des points de vue. Par ailleurs, dans un contexte de tensions sur les recrutements dans la filière nucléaire, tensions liées à la relance de cette dernière, cette évolution doit permettre de regrouper les compétences rares tout en améliorant l’attractivité de ses métiers, au travers d’une diversité des statuts possibles, des parcours de carrière, y compris sur le plan géographique, et par des mesures d’ordre salarial permettant d’engager un nécessaire rééquilibrage par rapport au secteur privé. J’en viens aux avancées apportées lors de l’examen de ce texte en commission, grâce à l’excellent travail mené par mes collègues rapporteurs, Pascal Martin et Patrick Chaize, dont je salue l’engagement. Je me réjouis de la consécration législative des groupes permanents d’experts, qui garantira une évaluation impartiale, ainsi qu’une prise de décision fondée fondée sur les meilleures pratiques et les connaissances les plus récentes. En outre, j’approuve l’inscription dans la loi du principe de publication des résultats d’expertise de l’ASNR, qui vaudra également pour les avis des groupes permanents d’experts, comme c’est le cas dans la pratique actuelle. La crédibilité du système de sûreté nucléaire repose sur cette exigence de transparence, absolument indispensable pour assurer l’acceptabilité de la relance de l’atome dans notre pays.

Le démantèlement de l’IRSN, qui a su démontrer historiquement sa rigueur et son indépendance, est en effet incompréhensible, sauf à imaginer que l’on souhaite ainsi affaiblir un contre pouvoir, capable d’apporter de l’objectivité dans le débat sur l’énergie nucléaire. au risque de vous surprendre, la répétition en boucle des termes « fluidification » et « simplification » pour justifier le démantèlement de l’IRSN n’a pas suffi à nous convaincre de son bien fondé. Ces mots sonnent creux, alors qu’il est reconnu, y compris à l’étranger, que notre organisation de sûreté nucléaire, reposant sur un système dual, fonctionne, même si elle pourrait, bien sûr, être améliorée. En outre, si très peu d’arguments en faveur de la fusion nous ont été présentés, la liste des risques générés par cette réforme est, quant à elle, très étayée. L’avis que la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement (CNDASPE) a rendu à la suite de la saisine que nous avions effectuée en février dernier est très clair : « Le moyen le plus sûr d’assurer la séparation de la gestion d’avec la recherche et l’expertise […] consiste à maintenir ces missions au sein de personnes morales différentes. » La tenue d’un dialogue tripartite entre EDF, l’ASN et l’IRSN permet une triangulation dans l’analyse de risque, ainsi qu’une diversité dans les points de vue, garante d’une anticipation et d’une meilleure analyse des enjeux liés aux décisions en matière de sûreté. Affaiblir ce système semble dangereux, alors que les catastrophes technologiques ont souvent, dans l’histoire, été liées à des problèmes organisationnels – cela a été clairement démontré par les chercheurs étudiant les accidents, que ce soit dans le domaine spatial, chimique, aéronautique ou nucléaire.

ces éléments donnent l’impression que ce texte est destiné à faciliter la relance à marche forcée du nucléaire, en affaiblissant les contre pouvoirs, quitte à ce que cela se fasse au détriment du niveau de sûreté. La mise en œuvre de cette réforme ne vient pas nous rassurer à cet égard, bien au contraire. Son calendrier, tout d’abord, est extrêmement rapide et semble à même d’entraîner de fortes désorganisations. Une entrée en vigueur au 1 janvier 2025 semble irréaliste, alors que l’on parle de relocaliser les quelque 1 700 collaborateurs de l’IRSN et de faire travailler ensemble des cultures différentes. Cette désorganisation arrive à un moment où l’activité de l’ASN et de l’IRSN augmente, sans garantie de renforcement des moyens humains, avec à la clé des conditions de travail fortement dégradées. L’intersyndicale de l’IRSN est d’ailleurs inquiète des conséquences de cette fusion pour les salariés ; elle alerte sur le niveau de sûreté qui pourrait en résulter. Car c’est l’attractivité de ces métiers, donc notre capacité à gérer le risque nucléaire, qui est en jeu. Autre point de forte inquiétude, la mise en place, au sein de la future Autorité, de la séparation entre expertise et décision, pilier fondamental de notre sûreté nucléaire, est insuffisante. Le texte n’apporte pas de garantie sur l’indépendance des experts, alors que l’IRSN était reconnu pour fournir des données de façon robuste et objective. Autres principes clés malmenés par ce texte, la transparence et le dialogue avec la société civile y sont en net recul par rapport au système existant. L’IRSN avait réussi à nouer un dialogue avec la société civile, et il est reconnu comme participant efficacement à la démocratie technique et environnementale. Rien n’indique que la future entité jouera ce rôle,quand la publicité de ses travaux n’est pas suffisamment garantie. Loin de la fluidité promise, cette réforme semble bancale et inaboutie, comme en témoigne le renvoi de nombreux points à un futur règlement intérieur,

par le Gouvernement. Nous sommes donc plus qu’inquiets, monsieur le ministre, face à cette volonté désormais très claire d’acter des retours en arrière sur la transparence et l’indépendance de l’expertise. Rappelons le, nous parlons ici de la sécurité de nos concitoyens et de notre environnement, non pas seulement pour aujourd’hui, mais pour des siècles Nous nous opposons à la relance nucléaire. Nous avons à maintes reprises souligné l’impasse financière et les risques liés à cette technologie. Mais, que l’on soit pour ou contre l’énergie atomique, la maîtrise du risque d’accident nucléaire reste une priorité et doit conditionner tous nos choix. Nous nous opposons donc plus que jamais à ce texte. Et si nous proposons des amendements pour tenter de limiter les risques qu’il comporte, nous vous appelons, mes chers collègues, à ne pas voter ce projet de loi : je le dis avec force,

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, pour les communistes, la relance et le développement de la filière nucléaire française doivent marcher sur deux pieds. En premier lieu, il faut un statut de haut niveau pour les salariés, y compris les sous traitants, qui reconnaisse leurs qualifications, avec un haut niveau de rémunération : un statut qui les protège et qui, donc, nous protège. En second lieu, il faut une transparence totale en termes de sûreté, pour permettre l’adhésion totale des citoyens et citoyennes, ainsi que des élus locaux. au moment où l’on s’apprête à relancer le nucléaire français, le Gouvernement décide dans le même temps de réformer le contrôle de sa sûreté. Très bien, mais dans quel but, et pourquoi ? Jusqu’alors, cette mission d’intérêt général reposait sur un système dual, composé de l’ASN, gendarme du nucléaire, et de son expert technique, l’IRSN. Ce système éprouvé n’a cessé d’évoluer pour garantir la conciliation entre une diversité de points de vue, ce qui a permis d’éviter le monolithisme décisionnel, vecteur de risques. Si des pistes d’amélioration sont toujours envisageables, le Gouvernement a fait le choix d’une restructuration dont le bien fondé a été très largement contesté par les personnels de l’IRSN et de l’ASN, mais aussi par de nombreux chercheurs et scientifiques. Aussi, monsieur le ministre, pourquoi défaire ce qui fonctionne ? Aucun des arguments que vous avez présentés ne tient la route. La vérité est donc ailleurs. Le Gouvernement, comme parfois l’exploitant, a toujours considéré que l’IRSN était un frein dans le développement du nucléaire et que, pour relancer ce secteur, il fallait y aller vite et fort – en réalité, en finir avec l’IRSN. Le résultat, c’est la désorganisation que nous constatons actuellement, principalement liée au fait que vous n’avez pas nommé de préfigurateur à la fusion et qu’il s’ensuit une grande incertitude, justifiée, chez les salariés de l’ASN comme de l’IRSN. Pour l’IRSN, près de la moitié de l’équipe de sécurité a démissionné. Il ne reste que trois personnes affectées au traitement des déchets radioactifs, et deux à la supervision des 56 réacteurs. Voilà les résultats de vos choix politiques : les salariés s’en vont déjà pouvez vous répondre à quelques questions simples ? Quels concours de recrutement seront prévus ? À quel niveau de rémunération ? Combien de postes seront ouverts ? Il faut que vous nous répondiez clairement sur vos ambitions pour assurer l’attractivité de cette nouvelle entité de sûreté nucléaire, d’autant que tous nos amendements ayant pour objet les salariés et la question sociale ont été déclarés irrecevables, ce qui est inacceptable.

Autre exemple, alors que la sûreté nucléaire militaire, jusqu’alors dévolue à l’IRSN au même titre que le nucléaire civil, risque d’être transférée au ministère des armées, des divergences d’avis de sûreté sont à craindre, en plus d’un recul sur la transparence. transparence. Pour les réacteurs SMR – une technologie transposée du domaine militaire au civil –, l’impossibilité de mobilités internes résultant de cette restructuration fera perdre des connaissances précieuses. Cela doit nous alerter, d’autant que ces nouveaux réacteurs seraient confiés à des acteurs privés, qui ne raisonnent qu’en termes de profit, et non d’intérêt général. Plus généralement, le présent projet de loi ne garantit pas le même degré d’indépendance et de sérénité de l’expertise. Or celle ci doit se fonder uniquement sur des faits scientifiques et rester hermétique à la faisabilité industrielle ou aux intérêts économiques et commerciaux. Actuellement, la production nucléaire est une activité hautement capitalistique. Les enjeux économiques liés aux décisions de démarrage ou d’arrêt des centrales sont donc prégnants. Si l’objectif de minimiser la durée d’exploitation, pour des raisons économiques, est compréhensible, nous considérons que l’impératif de sûreté doit toujours primer. Plus encore, ce projet ne garantit pas la pérennité des exigences actuelles en termes de transparence et de démocratie environnementale, alors que ce sont là des valeurs fondamentales, ainsi qu’un maillon essentiel de la confiance des citoyens et des citoyennes envers le secteur nucléaire. Si la publication des avis de l’IRSN reposait auparavant sur un fondement légal, le texte, tel qu’il nous est présenté, relègue cette possibilité, de manière vague, au domaine du règlement intérieur. Ainsi, contrairement à la communication gouvernementale, qui assure que ce projet de restructuration vise à renforcer et fluidifier le contrôle de la sûreté nucléaire, nombre des effets potentiels du texte semblent nous éloigner des objectifs annoncés. Pour toutes ces raisons,

beaucoup de mes collègues, à me forger une conviction solide quant à la pertinence du projet de loi qui nous est soumis. Ce n’est pas faute d’avoir cherché des arguments objectifs, au delà des clivages idéologiques.

Néanmoins, la relance historique de notre filière nucléaire exige que nous repensions et adaptions l’organisation de notre sûreté nucléaire. Il est possible que ce texte apporte une réponse concrète à cette obligation de membres du groupe RDSE le pensent. Quoi qu’il en soit, les débats qu’il suscite sont essentiels : faire la démonstration de la sûreté d’un système, c’est d’abord le confronter au doute

qui ont vécu des fusions de collectivités savent bien que le gigantisme n’est pas toujours synonyme d’efficacité, loin de là. Nul doute aussi que, derrière la fusion, se cachent des enjeux de gouvernance, qui mériteraient aussi d’être posés sur la table. Dans cette même logique de clarification, vous me permettrez de louer les travaux effectués par nos rapporteurs en commission. Ils ont cherché à préserver une distinction des responsabilités entre l’expertise et la décision, à renforcer l’expertise indépendante en consacrant l’existence des groupes permanents d’experts (GPE), à garantir un niveau de transparence élevé, à prévenir les conflits d’intérêts, notamment pour préserver les capacités de recherche, ainsi qu’à mieux associer le Parlement et la société civile. civile. Ces apports de la commission ne risquent ils pas, toutefois, de créer tout simplement un nouveau système bicéphale, une hydre à deux têtes ? le maintien de notre sûreté nucléaire au niveau d’exigence et de transparence le plus élevé possible, d’autre part ; mais cette fusion risque d’entraîner une désorganisation du fonctionnement de deux organismes qui ont appris, au fil des années, à travailler en bonne intelligence. intelligence. Le calendrier de ce projet de loi nous interpelle aussi. La fusion de différentes structures peut déboucher sur un travail d’intégration administrative qui est susceptible de durer des années. Avons nous des années à sacrifier à une telle réorganisation, alors que l’on parle de la mise en route des premiers réacteurs de type EPR2 à

Je pense à une augmentation substantielle des ressources de l’IRSN et de l’ASN, pour garantir leur soutenabilité sur le long terme, à la poursuite de l’effort d’augmentation des moyens humains de ces deux entités et à la révision de leurs politiques de ressources humaines, afin de renforcer l’attractivité de leurs métiers. Le nucléaire a un rôle clé à jouer dans la politique énergétique française du XXI siècle, pour renforcer la souveraineté de la France et pour répondre à l’exigence de disposer décarbonée, pilotable et disponible ! Notre contrôle de la sûreté nucléaire a permis de faire accepter cette énergie auprès de nos concitoyens. Je ne sais pas s’il faut prendre le risque de sacrifier cette confiance pour plus d’efficience.

faire de la France le premier des grands pays industriels à sortir de la dépendance aux énergies fossiles, tel est l’objectif fixé. Cela passera par la relance, historique, de notre filière nucléaire. Ce texte est donc primordial. Les deux tiers de notre consommation d’énergie finale émanent encore aujourd’hui des énergies fossiles. Nous devons accélérer la décarbonation de notre pays et développer la production massive d’énergie décarbonée, qu’elle soit nucléaire ou renouvelable. Nous partageons tous ici une ambition commune : remettre notre pays sur la bonne trajectoire énergétique. Si l’on attend avec impatience le projet de loi sur la souveraineté énergétique, l’objectif de la stratégie française pour l’énergie et le climat,

Cette stratégie exige donc que nous accélérions fortement le rythme sur les énergies renouvelables et sur le nucléaire, de façon continue et de façon structurelle. Je salue en ce sens la création d’une délégation de programme interministérielle au nouveau nucléaire, le déploiement de crédits d’investissement massifs dans le cadre des plans France Relance et France 2030, la tenue de conseils de politique nucléaire, ainsi que les victoires acquises par le volontarisme d’Agnès Pannier Runacher, telles que la nouvelle définition de la taxonomie verte et la création de l’Alliance du nucléaire, qui permettent de placer cette énergie au cœur des politiques européennes. Comme l’a souligné le Gouvernement ces derniers mois, la relance du nucléaire passera par la prolongation du parc existant, le développement de nouveaux réacteurs nucléaires français – les EPR2 et les SMR –, et par de nouvelles solutions de stockage des déchets. Alors que nous n’avons développé qu’un seul EPR depuis dix neuf ans, cette relance du nucléaire demandera une montée en charge et en capacité inédite pour la filière depuis le plan Messmer.

Afin d’assurer une pleine maîtrise industrielle et le maintien des standards de qualité et de sûreté au plus haut niveau imaginable, dans le contexte hors norme que nous connaissons et qui a été rappelé, le Gouvernement a fixé quatre objectifs qui constituent autant de principes qui devront guider l’examen de ce texte l’amélioration de l’efficience des procédures ; l’indépendance de l’autorité vis à vis des exploitants nucléaires et du Gouvernement ; l’exigence d’une transparence renforcée vis à vis du public ; et l’amélioration de l’attractivité des métiers, pour que la nouvelle autorité bénéficie de compétences et d’une expertise d’excellence.

l’accompagnement des changements majeurs dans les procédures de travail des 500 fonctionnaires et contractuels de droit public de l’ASN et des quelque 1 600 salariés de droit privé de l’IRSN, dans une configuration inédite pour une autorité administrative indépendante ; et, enfin, la mise en œuvre claire des dispositions sociales qui figurent dans le projet de loi. Notre commission a également créé, au sein de la future autorité, une commission d’éthique et de déontologie composée de personnes extérieures qualifiées, sur le modèle de celle qui existe actuellement pour l’IRSN.

nommés en raison de leurs compétences – les modalités de nomination seront précisées dans le règlement intérieur de l’autorité. Le groupe RDPI, vous l’avez compris, salue la plupart des évolutions intervenues en commission et se prononcera en faveur de ce texte. La parole

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, malgré le travail des rapporteurs, que je salue, ce projet d’intégration de l’IRSN dans l’ASN ne nous paraît pas suffisamment fondé en raison. Son étude d’impact, faible, ne définit pas clairement les objectifs. S’agit il d’aller plus vite ? De faire des économies ? D’améliorer les processus d’expertise et de décision ? On ne sait pas.

s’en est ému officiellement lors de sa séance du 25 janvier dernier. En résumé, on fait tout à l’envers depuis le début, et on persévère à chaque occasion ! On travaille au coup par coup, sans perspective d’ensemble. Ne croyez vous pas que le titre II de ce projet de loi aurait dû figurer, il y a des mois, dans la loi de relance du nucléaire ? Plus grave, la perspective du développement de petits réacteurs SMR, stratégique pour la décarbonation de l’industrie,

L’enjeu majeur, c’est de gagner la confiance de toutes les parties prenantes, dont le grand public. Or il n’y aura pas de confiance publique sans transparence totale. De surcroît, la question des moyens financiers nécessaires à l’augmentation de charge est renvoyée à un rapport. les perspectives d’exercice et d’évolution pour les métiers, hautement qualifiés, concernés ? Les personnels sont inquiets. Nous n’avons pas de réponses à toutes ces questions majeures. Nous n’avons pas non plus de proposition d’optimisation de l’organisation existante ni d’évaluation de cette dernière au regard des objectifs sont, il faut le reconnaître, peu ou pas formulés. Pour toutes ces raisons de fond, nous nous opposerons à ce projet de loi. Très bien… Cependant, en responsabilité et dans la continuité des échanges que nous avons eus avec l’Anccli et les et les syndicats des deux établissements, nous proposerons des amendements pour renforcer la sûreté et la radioprotection en France. La parole Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, les projets de loi que nous examinons actent la fusion de l’Autorité de sûreté nucléaire et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire au sein d’une autorité unique de sûreté nucléaire et de radioprotection. Ces textes visent à renforcer l’attractivité des métiers, à accroître la transparence du nouvel organisme vis à vis du public et à garantir l’efficience de la sûreté nucléaire. Bien que techniques, ces dispositions sont utiles et bienvenues pour accompagner la relance du programme nucléaire civil français que nous appelons de nos vœux depuis plusieurs années au Sénat. Elles s’inscrivent dans le prolongement de la loi sur l’accélération du nucléaire, que nous avons votée en juin dernier et qui doit permettre de revenir sur les erreurs fatales commises par le passé,

de l’examen en commission, les rapporteurs, que je salue, ont proposé un certain nombre d’ajustements, afin de fluidifier davantage encore les différentes procédures, notamment les règles de la commande publique concernant les projets de recherche, de production et de stockage nucléaires.

Si nous sommes nombreux à souscrire pleinement à cette réforme, je souhaite néanmoins insister sur un triple enjeu qui me paraît essentiel : la formation, la compétence et l’attractivité des métiers de la filière nucléaire. Cette réforme conforte les moyens humains de l’autorité de sûreté nucléaire, en la laissant plus libre de redistribuer ses ressources humaines entre les nouveaux projets nucléaires et le nucléaire historique.

Comme je le disais, nous voterons cette réforme, car la majorité sénatoriale défend depuis plusieurs années, avec force, la relance du nucléaire civil. En 2021, nous avions déjà adopté deux résolutions sur ce sujet et sur l’intégration de l’énergie nucléaire à la taxonomie verte européenne. mission d’information transpartisane sur l’énergie nucléaire et l’hydrogène bas carbone a également abondé en ce sens. Il s’agit à présent de tenir nos objectifs

C’est une étape nécessaire si nous voulons préserver notre indépendance énergétique, nous inscrire dans la lignée des plans Messmer, tout en agissant pour le climat, et ce dans l’intérêt bien sûr de nos concitoyens,

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le 30 janvier dernier, lors de sa déclaration de politique générale, le Premier ministre a rappelé le caractère crucial du nucléaire pour l’avenir énergétique de notre pays et son indépendance. Si nous voulons être à la hauteur de nos ambitions, nous devons agir à tous les étages de la fusée de l’atome, de l’industrialisation jusqu’à la supervision des activités, en passant par la formation, la recherche et l’innovation. Notre effort sera total ou ne sera pas. À ce titre, ces projets de loi constituent une étape qu’il nous faut saluer. Ils nous doteront d’une autorité moderne, aux moyens financiers, juridiques et humains adaptés aux enjeux contemporains. Ainsi, le groupe Union Centriste soutient ce projet de fusion de l’ASN et de l’IRSN, qui permettra de former la future ASNR. Frappée du coin du bon sens, cette réforme est la bienvenue. est la bienvenue. Je souhaite d’ailleurs saluer le travail réalisé par nos rapporteurs, Pascal Martin et Patrick Chaize, qui ont permis de corriger certaines malfaçons et d’enrichir ce texte. Nos lignes rouges ont été respectées. Tout d’abord, les salariés des deux entités bénéficieront des garanties liées à leurs différents statuts de droit public La diversité des parcours sera une force de l’institution. pour lancer les chantiers cruciaux du nucléaire, mais également sur une autorité de sûreté, capable de mettre l’expertise et la rigueur scientifique au cœur de son réacteur décisionnel. Malgré cela, des défis attendent la future autorité à commencer par la question de son attractivité : de l’ordre de de revenus entre les membres de la future ASNR et les salariés des entreprises privées. Cette réforme ne nous exonère pas de notre responsabilité face à ce problème qui perdure. Que proposez vous, monsieur le ministre, pour améliorer l’attractivité de ces métiers ? ne constitue pas le seul point de vigilance de notre groupe. En effet, si le texte va dans la bonne direction, la distinction entre les missions doit être inscrite dans notre droit et doit être respectée dans les faits. Nous devons pouvoir être les garants de cette indépendance grâce à un contrôle rigoureux. Il y va de la crédibilité des rapports de l’ASNR. Parallèlement, nous appelons de nos vœux un meilleur encadrement des relations de l’autorité avec les autres acteurs de l’écosystème nucléaire, à l’image d’EDF. Les impératifs économiques ne doivent pas prendre le pas sur la sûreté de nos installations. Enfin, le transfert de l’expertise nucléaire de défense au ministère des armées a tout de la fausse bonne idée. L’ASNR doit garder cette compétence dans son giron et s’appuyer si nécessaire sur l’expertise des services de l’État en matière de défense. Vous le voyez, monsieur le ministre, nous saluons la copie, mais la rédaction reste perfectible. La grammaire du nucléaire mérite des ajustements qui ne sont pas de l’ordre de l’anecdote. Le groupe UC y veillera. La parole

malgré aussi les campagnes de diabolisation des écologistes, malgré enfin l’abandon du démonstrateur Astrid ou encore la fermeture de Fessenheim. La filière nucléaire française doit renaître de ses cendres. Après de multiples tergiversations et atermoiements, et – il faut le dire – un revirement assez acrobatique, le Président de la République a enfin donné une direction, lors de son discours de Belfort en janvier 2022, faisant enfin du nucléaire la pierre angulaire de notre politique souveraine énergétique. Il était temps ! Le Parlement a, depuis, adopté la loi du 22 juin 2023. juin 2023. Nous examinerons bientôt le futur projet de loi relatif à la souveraineté énergétique, dont la déclinaison se fera au travers de la nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie et de la stratégie nationale bas carbone. Le nucléaire y aura enfin toute sa place ! Mais que de temps et de compétences perdus durant ces trente dernières années ! Et à quel prix ? Celui de la fragilisation de notre filière nucléaire d’excellence ou encore de l’importation d’électricité carbonée. Dans le cadre de la nouvelle donne, le Gouvernement prévoit donc une réorganisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire par le biais de la fusion de l’ASN et de l’IRSN. Le Gouvernement a bien essayé de passer en catimini, en déposant deux amendements à l’Assemblée nationale de l’examen du projet de loi sur l’accélération des procédures de construction de nouvelles installations nucléaires. Cette tentative a logiquement échoué, tant le Gouvernement avait bâclé son projet en ne menant pas en profondeur les consultations nécessaires pour permettre aux parlementaires d’avoir d’un avis éclairé. Fort opportunément, le Parlement a alors saisi l’Opecst réalise un vrai travail de fond sur les conséquences d’une éventuelle réorganisation de l’ASN et de l’IRSN. Nos collègues Fugit et Piednoir ont formulé des propositions visant à créer une grande autorité indépendante de la sûreté et de la radioprotection, dont les moyens financiers et humains seraient renforcés. Le Gouvernement a, pour sa part, mené une série de consultations auprès de différentes institutions. Ces débats n’ont donc pas été inutiles pour parvenir à l’élaboration d’un projet plus mature sur le fond.

notamment de renforcer les capacités d’expertise de la nouvelle entité. La future ASNR remplacera donc l’ASN et elle se verra attribuer les prérogatives de l’IRSN, qui est actuellement chargé d’effectuer des recherches sur les risques liés à la radioactivité. Récemment, le président de l’ASN a apporté son soutien à cette fusion clarificatrice. Il a souligné que le dispositif actuel n’a pas été conçu pour faire face à un contrôle de sûreté dans le « contexte hors norme » lié à la relance de la filière nucléaire française, notamment par la poursuite de l’exploitation des réacteurs existants, la réalisation de nouveaux réacteurs, le stockage géologique ou sur site du combustible, et la création d’installations de fabrication et de retraitement du combustible. Le texte vise ainsi à créer une organisation resserrée : institution d’un interlocuteur unique, unification du pilotage des priorités, regroupement des compétences, fluidité des processus d’instruction.

Le niveau de sûreté dépendra bien évidemment de l’efficience des procédures de contrôle. Comme le souligne le président de l’ASN, la réalisation de six EPR2 ainsi que le développement des réacteurs SMR () ou AMR () pourraient mettre en tension la chaîne d’approvisionnement de la filière nucléaire. une multiplication de contrefaçons, d’irrégularités ou de fraudes est alors à redouter. Il a rappelé aussi que le contrôle, à tous les niveaux de la chaîne, doit rester un point majeur de vigilance pour toute la filière.